Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chère Jocelyne Guidez, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de clore avec vous aujourd'hui le chapitre parlementaire concernant cette cette proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Je souhaite avant tout remercier chaleureusement son auteure, la sénatrice Valérie Létard, dont l'engagement et la maîtrise auront permis de mettre ce sujet sur la table, d'en faire un véritable objet politique et d'aboutir à un texte qui, rapidement, pourra produire de pleins et utiles effets. Je me permets également de saluer la présence en tribune de la députée Valérie Six,

Je sais que les habitants des régions les plus touchées par le phénomène d'usage détourné du protoxyde d'azote sont nombreux à attendre avec impatience l'entrée en vigueur de cette loi. À Tourcoing et dans d'autres villes, on ne connaît que trop bien les ravages que peut causer ce geste d'apparence anodine, qui consiste à aspirer une petite quantité de gaz issu d'un banal contenant.

Ce produit de consommation courante, utile à certains professionnels ou à certains cuisiniers amateurs, souffre aujourd'hui d'une bien mauvaise réputation. Il faut dire que la documentation est étoffée sur ses détournements. On l'a vu utilisé dans des bars, dans des soirées étudiantes, dans des fêtes foraines ; on l'a vu vendu par des buralistes ou facilement accessible sur internet, dans des emballages dont le marketing ne laissait pas de place au doute quant à l'usage qui en serait fait on a vu des mineurs en consommer, parfois encouragés par des adultes inconscients des risques ou à l'insouciance qui frôle la mise en danger d'autrui. Il était devenu insupportable pour les responsables politiques et pour les autorités sanitaires de constater une telle déconnexion entre les comportements des individus et les risques avérés. Je rappelle que le ministère de la santé avait publié deux communiqués de presse qui alertaient sur les risques liés à cet usage détourné, en novembre 2019 puis en juillet 2020, à l'occasion de la publication des données de l'Agence Une campagne d'information et de réduction des risques avait par ailleurs été lancée pour toucher directement non seulement les consommateurs, y compris les plus jeunes, mais aussi les acteurs de terrain : associations, collectivités locales, encadrants et personnes en lien avec les jeunes. Bien sûr, il fallait que cela s'accompagne d'un changement législatif. En ce sens, cette proposition de loi a été plus que bienvenue, à un moment important. Tout son parcours plaide d'ailleurs en sa faveur. Si le temps a pu paraître long depuis son premier examen, ici même au Sénat, la faute n'est pas à chercher, une fois n'est pas coutume, du côté d'éventuelles dissensions politiques. Les avis, au contraire, ont été très largement partagés sur l'opportunité d'avancer et, globalement, sur les termes des mesures à mettre en oeuvre. Sénat et Assemblée nationale ont chacun apporté leur contribution à ce texte, contribution que le Gouvernement a estimée parfaitement utile et cohérente

Parents, amis, équipes éducatives : toutes et tous doivent également en être informés. Cette prévention doit aussi se faire à l'égard d'autres produits, car les mésusages se déplacent régulièrement vers d'autres substances, par effet de mode ou du fait de l'interdiction d'une pratique Les pouvoirs publics sont et resteront pleinement mobilisés sur ces enjeux, autour du ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, et à travers un réseau puissant, structuré, notamment par les agences régionales de santé Je rappellerai, pour conclure, que des dispositifs d'aide sont à disposition des jeunes, de leurs entourages et du public en général, car la loi n'est jamais stigmatisante. Elle est faite avant tout pour protéger et accompagner les publics à risque. Il ne faut Il ne faut donc pas hésiter à se saisir de ces différents outils en cas de questions ou de difficultés liées à la consommation de produits ou de drogues. Je pense évidemment aux consultations jeunes consommateurs (CJC), qui proposent un service d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation. Ce service, assuré par des professionnels des addictions, est dédié aux jeunes ; il est entièrement gratuit et confidentiel. Je pense également à des dispositifs d'aide à distance,

c'est en agissant par cette pluralité de canaux que nous arriverons à véritablement protéger nos concitoyens de dangers, que, trop souvent, ils ignorent ou minimisent. Ne relâchons pas notre vigilance, à l'instar de Mme la sénatrice

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est en grande partie grâce à Valérie Létard que tout le monde le sait désormais : l'usage détourné du protoxyde d'azote à des fins récréatives est une pratique dangereuse, au succès inquiétant. Elle est d'autant plus dangereuse que ceux qui s'y livrent ignorent sa dangerosité, et son succès est d'autant plus inquiétant qu'il concerne essentiellement les mineurs et les jeunes majeurs. La proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ainsi que les députés l'ont rebaptisée, n'a jamais été si proche de son entrée en vigueur, et je suis convaincue qu'elle permettra de lutter efficacement contre ce fléau. D'abord, la vente de ce produit sera mieux encadrée, puisqu'elle sera interdite aux mineurs ainsi qu'aux majeurs dans les débits de boissons et les débits de tabac. La vente des ustensiles liés à l'usage récréatif du gaz sera également interdite, et une quantité maximale de vente aux particuliers sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la santé. Ensuite, la prévention sera renforcée par la mention obligatoire, sur les contenants du gaz, de la dangerosité de son usage détourné, et par le renforcement des modules de prévention aux conduites addictives organisés dans le cadre scolaire. Enfin, parce qu'il faut enrayer la propagation de ce qui est vu, bien à tort, comme un loisir anodin, la provocation d'un mineur à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, et plus largement de tout produit pour en obtenir des effets psychoactifs, sera pénalisée. Nous pouvons sans doute regretter que l'Assemblée nationale ait renoncé à la mise à contribution des intermédiaires numériques dans la prévention des usages dangereux en supprimant un article jugé ambigu. Nous pouvons aussi déplorer que le Gouvernement n'ait pas souhaité étendre le délit de provocation aux majeurs. Nous pourrions enfin désapprouver le fait que l'interdiction de vente n'ait pas été étendue aux stations-services, comme cela avait été proposé en séance publique par les députés, ou que la question de la consommation de protoxyde d'azote au volant n'ait pas été abordée. À cela s'opposaient des arguments juridiques, pratiques ou politiques, mais, au fond, ne dit-on pas que le mieux est l'ennemi du bien ? Pour bien faire, il est grand temps que ces premières dispositions s'appliquent. Ce texte a en effet été déposé au Sénat en avril 2019.

Il aura ainsi fallu plus de deux ans, mes chers collègues, pour que l'encadrement minimal d'un produit à la dangerosité avérée puisse entrer en vigueur. Il faudra encore un peu de temps avant que la Commission européenne ne donne son autorisation à de telles restrictions d'échange d'un produit de consommation courante. Cela se comprend, et je ne plaide assurément pas contre le temps de la réflexion parlementaire ; mais peut-être aurions-nous pu tirer plus tôt ou plus vite les conséquences qui s'imposaient de l'observation d'un phénomène de mode que les Britanniques, notamment, connaissent bien depuis de nombreuses années déjà. En attendant, l'usage récréatif de ce gaz est à présent devenu un segment comme un autre de l'économie des stupéfiants, avec ses grossistes avisés, ses intermédiaires spécialisés et son marketing agressif. Quoi qu'il en soit, ce texte permettra de lui porter les premiers coups. Réjouissons-nous que le Gouvernement se soit rangé à l'analyse clairvoyante de Valérie Létard ; remercions Valérie Six et nos collègues députés de leur remarquable contribution à l'efficacité du dispositif, et saluons le travail des élus locaux, Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la satisfaction l'emporte donc sur les regrets, mais c'est encore une satisfaction inquiète : alors que nous sortons péniblement d'une situation de crise sanitaire sans précédent, et que les alertes sur la santé mentale des jeunes se multiplient,

utilisé comme gaz de pressurisation d'aérosol alimentaire, le protoxyde d'azote, aux effets euphorisants, est aujourd'hui massivement utilisé comme drogue récréative par les jeunes. Cette nouvelle mode constitue un réel danger pour leur santé. L'évolution de ces pratiques s'accompagne, en effet, d'une augmentation du nombre de signalements d'effets sanitaires graves, avec des atteintes du système nerveux central et de la moelle épinière, comme l'ont souligné les experts de l'ANSM. L'Occitanie figure parmi les trois régions qui comptent le plus d'intoxications au gaz hilarant. L'été dernier, dans mon département de l'Hérault, des communes, en particulier littorales, ont connu durant la saison touristique une vague de violences graves et une hausse importante des incivilités, des comportements intolérables souvent causés par cet usage détourné du protoxyde d'azote. Un certain nombre de maires ont ainsi dû prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, des arrêtés municipaux interdisant l'utilisation de ce gaz dans l'espace public. Afin d'apporter une réponse concrète à cette réalité de terrain, qui alerte de plus en plus les acteurs locaux, élus, professionnels de la santé, mais aussi les forces de l'ordre, nous avons adopté à l'unanimité, le 11 décembre 2019, la proposition de loi présentée par notre excellente collègue Valérie Létard

d'interdire la vente de protoxyde d'azote par les sites de commerce électronique. D'autre part, je souhaitais que soit dispensée une information sur les risques pour la santé de son usage détourné dans les établissements scolaires. L'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi à l'unanimité le 25 mars dernier, preuve d'un large consensus sur ce sujet. Ce texte va donc modifier le code de la santé publique, en prévoyant que le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante, tel que le protoxyde d'azote, pour en obtenir des effets psychoactifs, sera désormais puni de 15 000 euros d'amende. De même, il sera interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. Les sites de commerce en ligne devront spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne. Par ailleurs, une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote sera apposée sur chaque unité de conditionnement. Je me félicite de ce que me félicite de ce que le texte conserve la mesure de renforcement de la prévention dans le cadre scolaire. L'information dispensée dans les établissements scolaires, déjà prévue pour la consommation de drogues, devra ainsi inclure les dangers de l'usage détourné du protoxyde d'azote. Enfin, à l'instar de Mme la rapporteure au nom de la commission, dont je tiens à saluer le travail, je regrette l'absence d'obligation d'information des internautes au moment de l'achat de ces produits.

Ce produit peut être acheté, pour une somme modique, par n'importe qui, en supermarché, bureau de tabac ou sur internet. Sa facilité d'accès, ajoutée à la publicité sur ses effets hilarants diffusée sur les réseaux sociaux, a popularisé son usage détourné comme un produit récréatif et festif chez des mineurs de plus en plus jeunes. Si la proposition de loi cible plus particulièrement les mineurs, la moyenne d'âge des consommateurs est de 21 ans. Sa consommation, souvent en groupe, peut aller jusqu'à 200 capsules par jour. Le gaz a une action immédiate et agit sur une courte durée. La plupart des consommateurs ignorent les conséquences de cette drogue, souvent prise en association avec de l'alcool ou d'autres stupéfiants. Les centres antipoison rapportent des risques d'asphyxie, de coma et d'atteintes neurologiques et neuromusculaires graves. Le principal problème est la facilité avec laquelle les jeunes consommateurs ont la possibilité procurer ce gaz en achetant des siphons à chantilly commercialisés librement en magasin et sur internet. En effet, son utilisation n'est soumise à aucune restriction, en dehors de quelques arrêtés municipaux dont la portée reste limitée. Le texte que nous examinons entend combler ce vide juridique pour protéger le jeune public des intoxications au protoxyde d'azote. Le coeur du texte vise à interdire la vente de gaz hilarant aux mineurs et à pénaliser l'incitation d'un mineur à en faire un usage détourné. Des éléments d'information sur la dangerosité du produit seront désormais obligatoirement visibles sur les emballages, ainsi que sur chaque siphon. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit une campagne de sensibilisation spécifique en milieu scolaire, étendue à l'ensemble des pratiques addictives. L'Assemblée nationale a contribué à enrichir les dispositions du texte en étendant l'interdiction de vendre du protoxyde d'azote aux mineurs à tous les lieux. Elle a aussi visé les ballons et les objets dédiés à cette consommation détournée. Ces dispositions vont permettre de protéger une partie des consommateurs des risques liés à la consommation de cette substance. Je rappellerai néanmoins que la moyenne d'âge des consommateurs est de 21 ans. Aussi, cette proposition de loi ne sera pas suffisante pour réduire les usages et prévenir les risques, notamment chez les jeunes majeurs. L'interdiction du produit se heurterait au droit européen, mais nous pouvons utilement limiter le nombre de cartouches que peut acheter un particulier, comme l'a fait le Danemark, confronté au même problème. Parallèlement, nous devons renforcer nos moyens de lutte contre le commerce illégal. Ces derniers mois, deux réseaux de trafic de gaz hilarant ont ainsi été démantelés en Seine-Saint-Denis. souligné en commission, la prévention des addictions reste un volet essentiel pour protéger les mineurs et les jeunes adultes de pratiques dangereuses. Elle doit se faire en lien avec les associations de terrain. Enfin, face au développement de la vente de produits stupéfiants sur les réseaux sociaux et sur les messageries privées, nous devons mettre en oeuvre un accompagnement à la parentalité à travers le numérique.

bien que centrée sur la prévention des usages dangereux du protoxyde d'azote, cette proposition de loi s'avère en fait générique et pourra s'appliquer à tout mésusage d'un produit de consommation courante pour la recherche d'effets psychoactifs.

inquiète les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les élus locaux, d'autant qu'il touche un public de plus en plus jeune. En 2018, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies nous alertait, car la consommation se banalisait, en parfaite méconnaissance des risques associés en matière de santé : effets immédiats, comme des pertes de connaissance, chutes ou asphyxies, et, en cas de consommation récurrente, des complications neurologiques ou des carences en vitamine B12.

Il n'est pas rare de voir des « bars à proto », où les jeunes achètent directement des ballons, à côté de débits de boissons. En février, le centre d'addictovigilance de Lyon et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes appelaient à une nouvelle campagne de sensibilisation sur les risques encourus par les jeunes consommateurs, ayant constaté « la [récente] recrudescence, au niveau de la métropole lyonnaise, des signalements d'atteinte neurologique, ainsi que la présence visible de bonbonnes dans l'espace public Pour le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues de Lyon, l'usage, installé depuis longtemps, est aujourd'hui plus fréquent. Originellement festif, il est devenu solitaire ou se fait en petit groupe, et les étudiants pris en charge étaient, pour la plupart, déjà consommateurs au lycée, voire au collège. Cette situation appelait donc une régulation. Tel est l'objet de ce texte. En encadrant la vente de ce gaz, y compris pour les publics majeurs, cette proposition de loi apporte une réponse aux élus locaux, démunis face à ce problème de santé publique. Il ne sera ainsi plus nécessaire que des maires prennent des arrêtés d'interdiction qui ne relevaient pas de leur compétence et qui, dès lors, ne pouvaient être efficaces. Néanmoins, précisons que les interdictions ne font pas tout. Le texte, heureusement, ne s'y limite pas. L'usage de ce produit n'est pas que ponctuel. Ainsi, chez certains s'est installée une véritable dépendance. D'ailleurs, la progression des signalements sanitaires durant la crise du covid-19 sonne comme une alerte sur une conduite devenue addictive pour une partie des usagers. Pour ceux-là, il est essentiel de traiter la relation qu'ils entretiennent avec le produit, au-delà du produit lui-même, qui peut être remplacé

Le Portugal, qui a décriminalisé en 2000 la consommation individuelle de toutes les drogues et privilégié l'accompagnement à la sanction, a obtenu des résultats concluants. Cette politique s'avère être un succès. Les associations de terrain appellent à multiplier les solutions de prévention et d'accompagnement des consommateurs, avec notamment la mise en place de structures spécialisées et un suivi social renforcé. Aussi, nous saluons l'équilibre de ce texte, qui appuie sur la prévention et l'information, l'étiquetage, et sur des actions de sensibilisation en milieu scolaire sur les risques de ces consommations. nous resterons attentifs aux moyens accordés à la politique de prévention et de réduction des risques. Considérant qu'il s'agit d'une réponse nécessaire et équilibrée à un problème de santé publique, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera ce texte.

Beaucoup de choses ont déjà été dites et je risque d'être dans la répétition. Le protoxyde d'azote est, à l'origine, un gaz à usage médical, utilisé pour ses propriétés analgésiques. Il sert également comme propulseur pour les siphons à chantilly. Ce produit bon marché est en vente libre sur internet et dans le commerce. Cependant, le protoxyde d'azote, ou N2O, est surtout connu de nos jeunes comme le « proto », un gaz hilarant à effet euphorisant. Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais d'un ballon, après avoir « craqué » la cartouche pour l'ouvrir. Malheureusement, cette consommation n'est pas sans risque : l'inhalation du protoxyde d'azote peut provoquer des brûlures, une asphyxie, voire une perte de connaissance, des intoxications, des effets cliniques, principalement neurologiques, allant jusqu'à des atteintes de la moelle épinière, mais aussi cardiaques et psychiatriques. L'arrêté du 17 août 2001 l'inscrit sur la liste I des substances vénéneuses ; il est ensuite soumis à une réglementation stricte par l'arrêté du 21 décembre 2001. Pour lutter contre ce fléau, les pouvoirs publics français pointent la nécessité de conduire des actions de sensibilisation. Actuellement, seul le détournement du protoxyde d'azote à usage médical est encadré par la loi. En revanche, celui à usage domestique n'est soumis à aucune restriction. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise à corriger ce vide juridique. Depuis 2017, de nombreuses petites cartouches grises contenant ce gaz sont retrouvées dans l'espace public, comme le souligne l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies dans son rapport publié en décembre 2018. Ce phénomène traduit une banalisation de sa consommation, qui, selon une étude de la mutuelle SMEREP, serait le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes. Les collectivités locales s'investissent déjà fortement dans la prévention. Par exemple, dans mon département de l'Eure, le maire de Vernon, François Ouzilleau, a pris en 2020 un arrêté municipal interdisant la vente ou le don de cartouche ou de tout autre récipient contenant du protoxyde d'azote à une personne mineure non accompagnée Une amende de 68 euros est prévue pour la détention, l'utilisation et le dépôt de cartouche dans l'espace public. Cela faisait plusieurs mois que la police municipale de Vernon, les services de la voirie et de la propreté urbaine constataient l'augmentation du nombre de cartouches au sol dans certains

Depuis juillet 2019, sous l'impulsion conjointe du ministère de la santé et de celui de l'éducation nationale, l'ensemble des collèges et lycées de France met progressivement en place des partenariats avec des consultations jeunes consommateurs, offrent aux jeunes et à leur entourage un service d'écoute et d'orientation totalement gratuit et confidentiel. Une campagne d'information de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) vise pour sa part à doter les acteurs de terrain- associations et collectivités locales -de supports de sensibilisation clairs et adaptés. La présente proposition de loi a aussi pour objet de renforcer la prévention et la meilleure information des jeunes fréquentant les établissements scolaires sur les risques de l'usage détourné du N2O.

souligne que le protoxyde d'azote représente, sous des airs légers, un véritable danger pour nos jeunes. Ce texte englobe l'ensemble des aspects d'une prévention efficiente efficiente et d'une dissuasion nécessaire pour protéger les mineurs. L'importance de cette proposition de loi est reconnue de tous ; plusieurs sénateurs de mon groupe et moi-même étions d'ailleurs cosignataires de ce texte.

sur cette situation ; certains d'entre eux ont pris des arrêtés interdisant la consommation ou la vente de protoxyde d'azote sur le territoire de leur commune, sans véritable effet. L'Assemblée nationale a souscrit à l'économie générale du texte et a décidé de maintenir en grande partie les éléments introduits par le Sénat ; avec le groupe du RDSE, je m'en réjouis. Elle a toutefois adopté plusieurs modifications à l'article 2, notamment en introduisant un plafonnement de la quantité maximale de protoxyde d'azote pouvant être vendue aux particuliers, plafond qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie. Cette mesure va certes dans le bon sens. Il convient toutefois de s'assurer que la restriction posée n'est pas excessive au regard de l'objectif recherché. Comme l'a rappelé notre rapporteure Jocelyne Guidez, cet arrêté ministériel ne pourra être pris qu'après avis de la Commission européenne. Le plafond sera par ailleurs déterminé au terme d'une réflexion conjointe

tout comme l'interdiction de la vente et de la distribution de tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en recevoir des effets psychoactifs. L'article 2 apporte en outre une clarification : c'est bien la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote et non l'usage du gaz en lui-même qui doit faire l'objet d'un étiquetage dédié sur chaque unité de conditionnement. En effet, dans des conditions normales d'utilisation, le gaz est employé à des usages médicaux, culinaires et industriels qu'il convient bien évidemment de préserver. Ce même article prévoit que la constatation des infractions aux interdictions de vente pourra être aussi réalisée par les agents de police municipale, les gardes champêtres, ainsi que les agents de surveillance de la Ville de Paris. Cette extension va dans le bon sens ; encore faut-il que les forces de l'ordre soient présentes en effectifs suffisants, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de nos territoires. L'article 2 permettait de renforcer les obligations applicables aux intermédiaires numériques d'informer sur les interdictions de vente aux mineurs de certains produits. Il a été supprimé par les députés. Nous le déplorons, car l'information et la responsabilisation des usagers restent, en matière de santé, les premières des priorités.

progrès. Cette proposition de loi constitue une belle avancée, que nous saluons sans réserve. Elle contribue à la sensibilisation des jeunes sur les conduites addictives ; elle permet d'informer sur la dangerosité de ce produit détourné de son usage ; elle punit la provocation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; enfin, elle interdit sa vente et son offre à des mineurs, dans les commerces physiques comme en ligne. Détourner un produit de consommation de son usage est une pratique qui ne concerne pas seulement le protoxyde d'azote. Malheureusement, l'innovation en la matière est sans limites Nous ne pouvons qu'appeler le Gouvernement à aller encore plus loin dans les domaines de la prévention, de l'aide à la parentalité et de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Pour l'heure, au regard de l'équilibre trouvé dans ce texte, le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi, avec enthousiasme et sans réserve.

du protoxyde d'azote, autrefois limité à certains milieux, notamment les facultés de médecine, est devenu une triste banalité : nombreuses sont les villes à voir des cartouches joncher les trottoirs. Ce phénomène touche particulièrement la région des Hauts-de-France, mais il concerne l'ensemble du territoire national et un public de plus en plus jeune. La consommation se banalise. Il nous faut donc, plus que jamais, alerter dès le plus jeune âge.

comme moi l'expérience d'effectuer une recherche sur internet ; quand j'ai tapé « gaz hilarant », une alerte publicitaire s'est affichée indiquant : « Oubliez les soirées ennuyeuses, essayez le gaz hilarant ! Livraison à domicile en 30 minutes ! Notre épicerie vous garantit une soirée pleine de fou rire ! Parmi les produits proposés, on trouve des tanks de 4 litres, pour 150 euros ! Alors, que pouvons-nous faire, en tant que parlementaires, face à ce détournement d'un produit de consommation alimentaire ? Notre collègue Valérie Létard, dont je tiens à saluer l'engagement sur ce sujet, a proposé d'agir en interdisant la vente de protoxyde d'azote aux mineurs et en créant un délit de provocation des mineurs Nous sommes favorables à ces mesures de répression si un équilibre est maintenu avec des mesures de prévention. Les mesures restrictives sont nécessaires, mais peuvent se révéler inefficaces si elles ne sont pas accompagnées d'une politique de prévention offensive. L'outil le plus efficace pour sensibiliser les jeunes sur les effets de cet usage du gaz hilarant demeure un discours de santé publique qui informe sur les risques posés par la consommation de ce gaz. faire appel à des jeunes formés sur les risques du protoxyde d'azote, qui iraient à la rencontre d'autres jeunes sur les lieux de consommation connus. Des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes, avec un message d'information sur les risques, sans stigmatisation : ce modèle a fait ses preuves, par exemple, C'est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de soutenir cette proposition de loi en créant, dès le prochain projet de loi de finances rectificative pour 2021, une ligne budgétaire venant financer une campagne nationale de prévention contre l'usage du protoxyde d'azote.

En conclusion, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera pour cette proposition de loi, comme nous l'avions fait en première lecture. La parole

le protoxyde d'azote est un problème. J'ai été très marqué par l'étude réalisée à l'université de Bordeaux auprès de plus de 10 000 étudiants : on y apprend que 13 % d'entre eux sont des consommateurs actifs

Des réseaux très bien organisés trouvent là une source de revenus bien moins risquée pénalement que le trafic d'autres substances.

notamment dans le domaine extrêmement important du lien de la politique des addictions avec la politique de santé mentale. Nous avons plusieurs fois, depuis un an, évoqué ce thème majeur et la nécessité de renforcer la politique de notre pays en la matière les dispositifs de santé mentale sont largement insuffisants et partiellement inopérants en matière de lutte contre les addictions. C'est une interrogation qui nous est adressée collectivement. Ainsi, quand je regarde la situation dans mon département de Paris, plus précisément dans le nord-est parisien,

sur les usagers de drogues présents dans la rue pour que le préfet de police décide de réagir et de déplacer les usagers de drogues dans un jardin public un peu plus loin. fait, tant que nous n'aurons pas ces dispositifs de santé mentale et d'accompagnement social, nous ne résoudrons rien du tout ! Je crains que la situation

donc pour ce premier pas énergique : nous voterons ce texte

cela, c'est du bon sens, c'est indispensable ! Ce travail est ce qui nous permet aujourd'hui de voter un texte qui, dans sa formule aboutie et définitive, offre une base législative adaptée à la prévention des comportements dangereux des mineurs

qui ont été autant de porte-voix et de défenseurs de ce texte. Aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes très heureux de vous retrouver et de nous dire que,

Dans les prochaines années, plus de 500 détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme islamo-djihadiste sortiront de prison.

Compte tenu de la particulière dangerosité et du risque élevé de récidive de la part de tels individus une fois leur peine d'emprisonnement accomplie, nous avions jugé nécessaire que des mesures de surveillance adaptées puissent leur être appliquées après leur sortie de détention. Dans sa décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le principe même d'une mesure de sûreté à l'égard de personnes condamnées pour terrorisme ayant purgé leur peine. Toutefois, en dépit

Malgré cette appréciation du juge constitutionnel, demeure l'impérieuse nécessité d'un dispositif permettant d'assurer le suivi de personnes qui, libérées à l'issue de leur peine, peuvent continuer à constituer une grave menace pour la sécurité publique.

Le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît, en conséquence, comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l'enjeu que représente, en termes de sécurité publique, la sortie de détention des condamnés terroristes, tout en offrant des garanties de réinsertion renforcées. Dans cette perspective, la présente proposition de loi, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, reprend le principe du dispositif adopté en juillet 2020- celui d'un suivi judiciaire prononcé au stade postsentenciel, d'une durée décorrélée des crédits de réduction de peine et d'un prononcé conditionné à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité appréciée en fin de peine tout en y apportant les aménagements destinés à le rendre pleinement compatible avec les motifs de cette décision.

En deuxième lieu, la proposition de loi exclut l'application de la mesure de sûreté aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Elle limite, par ailleurs, le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d'un sursis simple. En troisième lieu, le texte prévoit que la mesure ne pourra être prononcée que lorsque l'individu concerné aura pu suivre un programme de réinsertion en détention, à l'instar d'autres mesures de surveillance judiciaire existantes. En quatrième lieu, même si cette précision était sous-entendue dans la rédaction adoptée par le législateur, le texte dispose explicitement que le renouvellement de la mesure ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une évaluation établissant la dangerosité, sur la base d'éléments actuels et circonstanciés. enfin, la proposition de loi introduit une gradation dans le prononcé des obligations susceptibles d'être imposées à la personne sortant de détention, afin de garantir que ne seront prononcées que des obligations strictement nécessaires et proportionnées à sa situation personnelle. Ainsi, dans le cadre du dispositif prévu, la juridiction pourra imposer aux personnes concernées le suivi d'un certain nombre d'obligations déjà applicables dans le cadre d'autres mesures de suivi judiciaire et qui relèvent, pour la plupart, d'un suivi social et d'un accompagnement personnalisé à la réinsertion. En revanche, le prononcé des obligations les plus attentatoires aux libertés individuelles- obligation de pointage, interdiction de paraître dans certains lieux et interdiction de fréquenter certaines personnes -serait réservé aux personnes pour lesquelles les premières obligations se révéleraient insuffisantes,

a lieu en présence du détenu, assisté d'un avocat ; une décision est prise. La mesure de sûreté ne peut être prononcée si le détenu n'a pu suivre un parcours de réinsertion ou des activités de réinsertion lors

monsieur le ministre,

votre travail. Ce texte s'inscrit pleinement dans l'objectif que s'est fixé le Gouvernement, celui de réduire au maximum une menace nouvelle et terrifiante : la possible récidive des personnes condamnées pour des actes de terrorisme qui, alors

des moyens sans précédent pour renforcer la réponse de nos services de sécurité et équiper la justice de tous les outils nécessaires au traitement de cette menace. Dois-je rappeler la création de 10 000 postes supplémentaires de gendarmes et de policiers, l'augmentation du budget de la justice, la création du parquet national antiterroriste, l'augmentation du nombre de quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER), l'augmentation du personnel affecté au renseignement pénitentiaire

J'ai, à cet instant, une pensée appuyée pour toutes les victimes des actes de terrorisme qui ont endeuillé notre pays.

d'ici à la fin de l'année 2024, 163 personnes actuellement détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste auront purgé leur peine. certaines d'entre elles présentent et présenteront sans doute encore des signes de radicalisation. série d'actions terroristes, le régime d'aménagement de peine en matière de terrorisme a été durci afin de répondre à la crainte que des personnes radicalisées et potentiellement dangereuses

Je tiens ici à saluer avec force l'important travail réalisé dans nos établissements pénitentiaires pour prévenir la radicalisation des détenus et de freiner tout prosélytisme délétère. Les services de mon ministère travaillent sans répit pour améliorer l'évaluation et la prise en charge des personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou présentant des signes de radicalisation.

121 places sur le plan national et un quartier réservé aux femmes incarcérées ouvrira à la fin de l'année 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes. nous disposons de 188 places de quartiers de prise en charge de la radicalisation à l'échelon national. Les détenus évalués comme étant en capacité de se soumettre à une prise en charge y bénéficient de programmes de désengagement, grâce à l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire, composée de médiateurs du fait religieux, de psychologues et de personnels pénitentiaires. Un quartier de ce type, réservé aux femmes détenues, ouvrira dans le courant de l'été 2021 au centre pénitentiaire de Rennes. Enfin, le Service national du renseignement pénitentiaire, dont nous avons augmenté les effectifs de 100 personnes en trois ans, assure un suivi très poussé de ces condamnés à leur libération, en lien très étroit avec les services partenaires du renseignement. du renseignement. C'est un constat partagé : la remise en liberté de détenus condamnés pour des faits de nature terroriste, potentiellement toujours radicalisés en dépit du travail réalisé, appelle une réponse forte et efficace. Il est de notre devoir de mettre tout en oeuvre pour garantir, dans le respect de notre État de droit, la sécurité de nos concitoyens. Le Gouvernement s'y est déjà attaché dans le cadre du dispositif issu de la loi SILT du 30 octobre 2017,

Pour autant, les conditions de la soumission à un nouveau régime judiciaire restrictif de liberté des personnes qui ont déjà purgé leur peine doit appeler à la plus grande vigilance.

s'inscrivait déjà dans la volonté commune qui nous réunit aujourd'hui d'apporter une solution à la nouvelle menace des sortants de prison condamnés pour terrorisme. Si, à la suite de cette censure, le travail il ne nous paraît pas suffisant pour parer à toutes les critiques alors formulées par le Conseil constitutionnel. Il ne saurait en effet être question d'instaurer ou de laisser penser que nous sommes prêts à instaurer une quelconque forme de justice prédictive : celle-ci est la négation de l'idée même de justice puisqu'elle revient à condamner sur un simple soupçon. Le respect de nos valeurs impose, à mon sens, que le régime applicable aux détenus terroristes

Celle-ci permettra d'assujettir le condamné à un suivi au moyen d'obligations et d'interdictions à vocation essentiellement sociale. Le projet défendu par le Gouvernement, qui sera bientôt examiné au Sénat, assure l'articulation entre le dispositif administratif-

certaines des obligations et interdictions auxquelles peuvent être astreintes les personnes concernées sont similaires ou voisines de celles qui sont prévues par les Micas, comme l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes. Une telle superposition paraît de nature à fragiliser la légalité des Micas prononcées à l'encontre des mêmes personnes, alors que ces mesures permettent précisément le prononcé d'obligations plus rigoureuses encore. D'une manière générale, le Gouvernement considère que la superposition de dispositifs de sûreté différents, sous la responsabilité d'autorités différentes, susceptibles d'être appliqués à des mêmes fins et aux mêmes personnes, en prévoyant des prescriptions similaires ou identiques, crée une complexité qui nuit à l'efficacité de l'action de l'État pris dans ses fonctions administratives et judiciaires. il convient de rappeler que les mesures de sûreté doivent respecter le principe résultant de l'article IX de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Comme je l'ai indiqué, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 août 2020, a rappelé la vigilance qui doit être celle du législateur sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de mesures restrictives de liberté lorsqu'elles sont imposées à des personnes ayant purgé leur peine. Or, précisément, certaines des dispositions de la présente proposition de loi, en particulier les conditions de renouvellement de la mesure de sûreté, ne semblent pas répondre aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel. Elles laissent craindre laissent craindre une nouvelle censure, qui doit absolument être évitée pour qu'enfin puisse être mis en place le nécessaire suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme. terrorisme. Nous sommes juridiquement sur une ligne de crête. Il appartient ainsi au législateur de prendre des mesures qui permettent d'assurer la protection des Français,

je ne peux, mesdames, messieurs les sénateurs, que saluer l'objectif de cette proposition de loi en ce qu'il rejoint l'engagement du Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme ; il confirme la détermination du Sénat en la matière. Je luis préfère toutefois

Les faits sont simples : 469 personnes sont actuellement détenues dans les prisons françaises pour des actes de terrorisme islamiste ; 253 sont condamnées et purgent leur peine 163 devraient être libérées dans les quatre prochaines années et présentent un risque réel de réitération des faits. Je crois important de revenir sur ces chiffres, qui figurent dans le rapport de Muriel Jourda. Ce risque n'est pas théorique : de trop nombreux attentats ont été commis sur notre sol, jusque dans nos centres pénitentiaires. La question des sortants de prison illustre de façon emblématique l'évolution d'une menace de plus en plus endogène dans notre pays. Nous éprouvons « plus qu'une inquiétude, une vraie peur » s'agissant « des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues. Elles constituent la menace prioritaire aujourd'hui ». Ainsi s'exprime Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste. Son constat est partagé par tous les acteurs concernés et nous dit l'urgence d'agir pour mieux protéger les Français. Aussi, le 27 juillet dernier a été adoptée la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine. En effet, la remise en liberté de détenus condamnés, potentiellement toujours radicalisés en dépit de l'accomplissement de leur peine et du travail réalisé, appelle des mesures spécifiques afin de prévenir la récidive. Il est donc de notre devoir de mettre tout en oeuvre pour garantir la sûreté de nos concitoyens. Dans sa décision du 7 août dernier, le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que le dispositif retenu par le Parlement portait une atteinte qui n'était ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Plusieurs articles de la loi ont été jugés contraires à la Constitution. En dépit de cette censure, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le principe de la mesure de sûreté. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi est essentielle. En effet, elle répond à l'enjeu que représente la sortie de détention de ces personnes qui ne bénéficieront pas de mesures d'accompagnement. Tout en reprenant le principe du dispositif adopté par le Parlement au mois de juillet dernier, ce texte y apporte des aménagements qui prennent en compte les objections formulées par le Conseil constitutionnel.

Je pense aussi à l'ajout d'un avis systématique du juge de l'application des peines pour éclairer utilement les décisions prises dans le cadre des mesures de sûreté.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les Français attendent de l'État qu'il les protège et c'est bien normal. La sécurité est l'un des fondements de notre contrat social. Si une menace existe, elle doit être prise en compte ; s'il existe un vide juridique, il doit être comblé. Tel est l'objectif de ce texte. Le combat contre le terrorisme est aussi et surtout un combat collectif : il exige la mobilisation de chacun- services de renseignement, forces de sécurité, magistrats et responsables politiques.

la sécurité des Français et l'intégrité du territoire national sont des préoccupations communes à tous les membres de la Haute Assemblée, je puis l'affirmer sans grande crainte.

On pourrait la résumer ainsi : toujours plus de répression judiciaire et pas assez de réflexion quant aux causes des problèmes que l'on entend traiter. En effet, le premier écueil de cette proposition de loi est d'ignorer la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent lors de leur détention. Il convient d'objectiver le phénomène de radicalisation en prison et de mettre en oeuvre un programme de réinsertion adapté et stable à ce type d'individus, pour qu'ils ne se retrouvent pas sans aucun accompagnement à la fin de la détention. Ensuite, cette proposition de loi ne pousse pas plus avant la réflexion sur les pratiques sociojudiciaires en matière de réintégration en milieu ouvert ou semi-ouvert des personnes radicalisées. se contente de mettre en place des dispositifs judiciaires de suivi de ces personnes. C'est tout le système de suivi des radicalisés qu'il nous faut peut-être revoir. Aujourd'hui, la stratégie de la France est celle du

Celle-ci implique des modifications du système de croyances conduisant à rejeter l'idéologie extrémiste au profit de nouvelles valeurs. Toutefois, elle est réductrice, car il s'agit encore une fois d'une approche confrontationnelle, qui porte difficilement ses fruits. Peut-être devrions-nous envisager de faire évoluer la conception de la prise en charge de ces personnes en France vers la notion de désengagement, qui, elle, s'inscrit dans la perspective d'un renoncement à la violence. Le Danemark a été un précurseur en la matière : dès 2007, il a employé une méthode basée sur le tutorat et l'accompagnement pour faire face à la radicalisation. extrémistes », ou RIVE, expérience inédite pour tenter de gérer la réinsertion des personnes radicalisées et leur suivi sous le contrôle des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Comment les individus sortis de prison perçoivent-ils leur propre réintégration ? Quelle est l'importance de l'implication des familles, des proches, des communautés dans la réintégration ? Comment les professionnels du travail social, de la justice et de la police adaptent-ils leurs outils et leurs pratiques à l'hétérogénéité des trajectoires et des besoins ? à l'heure actuelle, peu de travaux portent sur la situation française permettant de croiser ces différentes dimensions dans l'analyse du processus de réintégration. Or il s'agit bien là d'un enjeu social et scientifique majeur. Ce texte est donc une occasion manquée de faire évoluer la stratégie de suivi des condamnés pour terrorisme à la sortie de détention. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre. La parole

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire de l'adaptation de notre droit pénal à une criminalité particulière. C'est une histoire à épisodes. Avec l'aggravation de la criminalité terroriste, qui commence en 2012 dans notre pays et, bien vite, dans le reste de l'Europe, notre législation se renforce à la fois pour mieux caractériser et rendre punissables les crimes et délits qui constituent ce mouvement pour adapter les procédures en prévenant les risques de prolongation excessive des jugements comme, il faut bien dire, le risque de l'intimidation de ceux qui instruisent et de ceux qui sanctionnent. Les règles de ce droit rénové, qui vise à combattre le terrorisme, sont maintenant à l'oeuvre. Le moment est opportun pour affirmer notre respect et notre soutien

à mesure que ce dispositif répressif s'est déployé, un problème est apparu qui surplombe notre discussion d'aujourd'hui : l'idéologie meurtrière qui a conduit à l'acte terroriste, notamment pour ceux qui sont condamnés pour complicité

la disponibilité mentale et la capacité de retour dans la norme, qui en sont la première condition. La dangerosité des anciens condamnés qui subsiste nous adresse une sorte de double défi rester fidèles aux principes d'une justice humaniste, écarter la menace vitale d'individus restant enclins à combattre la société par le meurtre. nous avons adopté une loi habilitant le juge à prendre, après l'exécution de la peine, un ensemble de mesures de sûreté à l'encontre des anciens condamnés pour terrorisme, dans le but de prévenir et, déjà, de détecter les agissements qui révéleraient leur tendance à vouloir de nouveau attenter au sort de nos concitoyens. Le Conseil constitutionnel a déclaré cet ensemble de mesures

Pourtant, cette loi avait reçu l'approbation des deux assemblées, avec une majorité assez large dans les deux cas et après un travail approfondi de leurs commissions des lois Beaucoup d'entre nous s'y étaient associés et je m'étais personnellement réjoui de vous entendre, monsieur le garde des sceaux, peu après votre entrée en fonction, apporter votre appui à ce dispositif. À présent, il faut reprendre la plume, puisque, d'une part, le risque à combattre est toujours aussi présent et que, d'autre part, le Conseil constitutionnel a au moins reconnu- j'appelle aussi votre attention sur ce point, monsieur le garde des sceaux -la conformité au droit constitutionnel de mesures individuelles de sûreté en pareille situation. Il est donc souhaitable d'adapter un système de suivi sous le contrôle du juge judiciaire et d'une rigueur moins serrée que la panoplie trop large que nous avions fixée l'été dernier.

Nous trouvons ce dispositif équilibré et adapté au danger qu'il faut combattre et nous espérons, rationnellement, qu'il sera cette fois jugé conforme aux exigences supérieures du droit.

pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste, parmi lesquelles un nombre significatif devrait sortir de détention ces prochaines années. Notre société fait donc face à un double défi part, celui de la réinsertion d'individus ayant déjà fait acte de leur dangerosité, de leur radicalité et du rejet de notre société ; d'autre part, celui de parvenir à les réinsérer sans renier la philosophie de notre État de droit,

Il a été rappelé les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a été contraint d'en censurer des éléments principaux, considérant qu'en l'état étaient imposées des obligations et interdictions portant une atteinte trop importante à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, nous nous réjouissons que le Conseil constitutionnel n'ait pas rejeté le principe de la mise en place de cette mesure. Il nous revient donc de trouver l'équilibre et la justesse qui permettront à ce mécanisme d'être définitivement adopté dans le respect de nos principes essentiels et tout en conservant l'espoir d'une efficacité en vue de la réinsertion des personnes condamnées pour des actes de terrorisme. Aussi les ajustements proposés par les auteurs de cette proposition de loi paraissent-ils de nature à satisfaire ces diverses exigences. Qu'il s'agisse de la durée de la mesure ou bien de l'encadrement des possibilités de cumul avec les mesures de sursis, ces éléments devraient permettre au dispositif de passer le stade du contrôle de constitutionnalité d'entrer en vigueur le plus tôt possible. De la même façon, je salue les ajustements répondant à la nécessité d'éléments nouveaux et complémentaires pour le renouvellement de la mesure de suivi. La censure constitutionnelle aura ainsi permis d'introduire une nouvelle évaluation établissant la dangerosité sur la base d'éléments actuels et circonstanciés. Il en va de même de la gradation introduite dans le prononcé des obligations susceptibles d'être imposées. J'ai l'espoir, à l'image de la position de la commission des lois, que la réponse apportée par cette proposition de loi sera de nature à permettre la constitutionnalité du dispositif, lequel prendra mieux en compte la situation, la personnalité ou le niveau de dangerosité de la personne visée par la mesure. la mesure. Je souligne enfin un point particulier. Cette proposition de loi intègre le principe suivant lequel la mesure de sûreté ne peut intervenir à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement que si la personne a pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Cela est évidemment bienvenu et nous permet d'aborder un sujet fondamental, celui du rôle de l'institution carcérale dans notre société. En effet, je crains qu'il ne faille voir ici l'aveu d'une forme d'échec. Et comment ! Certes, la prison punit, mais elle ne prépare pas suffisamment à la sortie. Elle joue son rôle de répression, mais ne prépare pas efficacement à la réinsertion, alors même que ce devrait être son rôle principal. De cette manière, nous en sommes réduits à une forme de fuite en avant : après les peines, nous voilà à instituer des mesures post-carcérales avec l'espoir qu'elles seront efficaces, alors même que la Qu'adviendra-t-il si celles-ci se révélaient à leur tour inefficaces ? Faudra-t-il travailler sur un nouveau dispositif qui permettrait un suivi encore plus étendu à l'issue de ces mesures ? Ce n'est évidemment pas la solution, mais cela nous alerte sur une forme de précarité face à laquelle nous devrons nous montrer vigilants dans les années à venir. Ce dernier point n'empêchera toutefois pas le groupe du RDSE de voter en faveur de cette proposition de loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 21 juillet 2020 a été discutée au Sénat la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté

Dans sa décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif retenu portait, en l'état de sa rédaction, une attaque qui n'était ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. les auteurs et défenseurs des propositions de loi initiales continuent à considérer que les mesures de police administrative, notamment les Micas, aujourd'hui privilégiées par les autorités pour assurer le suivi des personnes libérées, représentent toujours une menace grave pour la sécurité publique et n'offrent pas un cadre de surveillance suffisant. Aussi proposent-ils de nouveau un renforcement du suivi judiciaire en proposant des garanties de réinsertion renforcées.

Rappelons que, lors de l'adoption de la rétention de sûreté, le sénateur Robert Badinter avait dénoncé « une période sombre » pour la justice. Il avait insisté sur « le brouillard » dans lequel cette « détention pour dangerosité, hors toute commission d'infraction », allait plonger la justice dont les fondements étaient atteints. Ces mesures induisent un bouleversement de la logique même du droit pénal. En effet, les mesures de sûreté ne sont pas relatives à une infraction commise. Elles ne visent que les « états dangereux Il n'existe donc pas de faute, le but de ces mesures étant seulement de protéger la société par des dispositions spécifiques permettant ainsi d'éviter notamment la récidive. On parle donc non pas de punition, mais de prévention. Il s'agit notamment- et dans la plupart des cas -d'utiliser ce genre de procédure pour réadapter des délinquants à la société par le biais d'une cure de désintoxication ou d'un internement, ce qui pose déjà grandement question. Présentées comme de simples moyens prophylactiques, ces mesures peuvent présenter un danger de dérive totalitaire. Or, en adaptant les mesures de sûreté aux personnes condamnées pour des actes terroristes, quel message envoyons-nous ? En pointant avec force la récidive probable, on envoie aux condamnés qui ont purgé leur peine le signal qu'ils sont suspectés à vie et, en quelque sorte, rejetés de la République. Ne nous leurrons pas : cette justice d'exception ne se bornera pas au seul cas des détenus terroristes, elle fera tache d'huile. N'est-ce pas déjà le cas au regard des lois votées à l'encontre des auteurs de délits et crimes sexuels, par exemple ? Pourtant, en creux, ce que révèlent notamment les mesures proposées, ce sont l'échec du temps pénitentiaire et l'épuisement d'un système basé sur le tout carcéral. Les vraies questions auxquelles cette proposition de loi ne répond pas sont nombreuses : quels moyens pour nos services de renseignements pour prévenir les actes de terrorisme ? Comment réinsérer dans notre société des individus condamnés pour de tels faits ? Les obliger, pendant plusieurs années, à se rendre jusqu'à trois fois par semaine dans un commissariat pour justifier de leur présence est un obstacle évident à la reprise d'une vie active et socialisante.

s'il ne serait pas sage, un an avant l'élection présidentielle, de sanctuariser au maximum notre code pénal. Quoi qu'il en soit, nous nous opposerons de nouveau à ce texte, qui continue, selon nous, malgré des aménagements à la marge, à aller à l'encontre des principes fondamentaux de notre État de droit, en instaurant en substance une peine après la peine. Comment faire

pour la prévention. À ce stade, je tiens évidemment à rendre hommage à nos services de sécurité, aux services pénitentiaires, aux services de renseignement, qui accomplissent un travail tout à fait remarquable, mais en aval.

ces établissements n'ont déjà pas les moyens de prendre soin de leurs malades. On a psychiatrisé le terrorisme avec des effets en cascade : des terroristes dangereux plongés dans le bouillon carcéral sortent plus délinquants qu'ils ne sont entrés. Les médecins experts, peu nombreux, ne peuvent jouer leur rôle.

? L'enjeu est majeur, mais nous ne pensons pas que cette proposition de loi, très proche finalement de celle qui a été censurée l'été dernier, soit la bonne réponse.

et les mesures préventives : il ne doit pas y avoir de mélange de responsabilités en matière de prévention des actes et en matière d'instruction sur les infractions et les crimes commis.

ceux qui luttent contre le terrorisme, en France et à l'étranger, dans la police, l'armée, la gendarmerie ou les services, dans la magistrature ou l'administration pénitentiaire, au nom du respect du rôle de chacun. Nous les devons aussi aux Français, au nom de leur sécurité. C'est pourquoi nous sommes opposés à cette proposition de loi, tout en sachant

Ravier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 62 condamnés pour des crimes ou délits terroristes islamistes sortiront des prisons françaises à l'issue de leur peine en 2021. Aujourd'hui, en France, il y a 469 personnes détenues en lien avec la mouvance islamiste, dont 162 qui seront remises en liberté dans les quatre prochaines années. Ces chiffres font froid dans le dos quand on sait à quel point certains de ces individus, que d'aucuns ont pu qualifier de « chances pour la France », demeurent endoctrinés, haineux et imperméables à toute réinsertion sociale. De véritables bombes à retardement que notre modèle juridique est incapable de désamorcer ! Le risque de récidive est sous-estimé, parce que nous ne sommes qu'au début du processus de libération de ces ennemis de la France. Que notre code pénal puisse donner les moyens à la justice de mettre hors d'état de nuire ces fanatiques, cela devrait être une évidence. Or, nous étions déjà là, il y a moins d'un an, pour débattre des mesures de suivi des terroristes sortis de prison. Nous y voici de nouveau, après censure du Conseil constitutionnel pour atteinte à certaines libertés fondamentales ! Les libertés fondamentales accordées à des fondamentalistes de la haine des libertés ... Cela ressemble à une mauvaise plaisanterie. De toute évidence, et d'expérience, on fait moins de cas des restrictions de liberté imposées par ce gouvernement aux honnêtes citoyens qu'aux ennemis de la Nation, coupables d'avoir financé des meurtres de masse, d'en avoir perpétrés, d'en avoir fait l'apologie, ou d'avoir tenté de rejoindre le théâtre d'opérations de pays en guerre. Ils bénéficient, eux, d'une protection juridictionnelle constitutionnelle. Les familles des victimes passées et à venir apprécieront ... La première des libertés, c'est la sécurité. Or, la sécurité des Français exige des restrictions de liberté à l'encontre de ceux qui leur ont déclaré la guerre. Débarrassons-nous de ces métastases du terrorisme, notamment par des mesures de déchéance de nationalité pour les binationaux, et d'expulsion pour les étrangers qui se seraient rendus coupables d'actes terroristes ou de complicité. On nous a souvent dit par ailleurs que les auteurs d'actes terroristes ou de menaces islamistes étaient des malades ou des déséquilibrés.

pas uniquement les outils juridiques. Quoi qu'il en soit, il ne servira à rien d'étendre perpétuellement les mesures de sûreté et de suivi des condamnés terroristes sortant de détention sans lutter efficacement contre l'origine de ce phénomène, dont la cause principale est l'immigration de masse, qui entraîne le communautarisme, lui-même terreau de l'islamisme. Combattons sans faiblesse les influences étrangères, les relais islamo-gauchistes, l'islam politique affiché ou dissimulé ! Restaurons l'autorité de l'État et réapprenons à être fiers de notre pays, de son histoire, de son identité. Il convient, mes chers collègues, d'ajouter aux solutions techniques et juridiques une vision, une action politique globale et déterminée reposant sur un postulat : la sécurité des Français avant les libertés des ennemis de la France

Nous sommes loin, si loin, de cette époque où tous les responsables agissaient en harmonie pour combattre l'insécurité. Ce regretté ministre de l'intérieur disait aussi que l'insécurité devait changer de camp et que, entre nous et les terroristes, la guerre était engagée. Oui, l'insécurité doit changer de camp ! Oui, il faut relever la police que l'on a mise à terre. Elle peut, soyez-en assurés, mes chers collègues, se tenir définitivement debout contre les terroristes, à condition de lui en donner les moyens légaux.

Instaurer une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance postsentencielle visant à prévenir la récidive et à accompagner la réinsertion des individus condamnés pour des faits de terrorisme est une nécessité absolue. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres, Sur les 269 condamnés pour terrorisme en lien avec la mouvance islamique suivis par le service de l'application des peines, 20 % seront suivis à leur libération dans le cadre sociojudiciaire, et 5 % dans le cadre d'un sursis probatoire. que 75 % d'entre eux pourront bénéficier de mesures d'accompagnement sur la durée des réductions de peine éventuellement octroyées. Le 27 juillet 2020, le Parlement adoptait une loi introduisant une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance postsentencielle

à notre arsenal judiciaire pour lutter contre le fléau que représente la sortie de détention des terroristes. La seconde est républicaine. Je veux lancer un appel, un cri d'alarme au Président de la République, aux ministres et à vous tous, mes chers collègues.

en France. Nous y sommes tous ici profondément attachés ; nous le respectons, il coule dans nos veines. Mais, aujourd'hui, n'en avons-nous pas une conception obsolète et naïve, qui coûte des vies ? Régulièrement, le Conseil constitutionnel censure des lois qui n'ont rien d'excessif et qui auraient pu sauver des vies, parce qu'elles sont en adéquation avec l'extrême violence qui prospère sans conteste dans notre société. Je vous le dis haut et fort, mes chers collègues, la loi doit être conforme à la Constitution,

proposer un référendum dont le seul objet serait d'ajouter le mot « développement durable » dans notre Constitution est superfétatoire. Ayez l'ambition et le courage de proposer un vrai référendum, un référendum utile pour la France et les Français, un référendum qui porte sur les moyens donnés à nos forces de sécurité et à notre système pénal pour lutter efficacement contre le terrorisme. L'urgence est indéniable ! La parole est à M.

de condamnés pour des faits de terrorisme constitue l'un des principaux enjeux sécuritaires d'aujourd'hui. En effet, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, ce ne sont pas moins de 162 détenus qui devraient être libérés dans les quatre prochaines années,

Certains de ces détenus sont probablement dangereux, et leur séjour en prison n'a sans doute nullement permis de mettre fin à leur engagement terroriste. nous n'avons pas la possibilité, alors qu'une peine a été prononcée et purgée, de prononcer une nouvelle peine pour les mêmes faits ; c'est la règle, qui est un principe fondamental de notre de notre code pénal. Aussi, la protection de la société ne peut être recherchée que par des mesures de surveillance et d'accompagnement, qui peuvent comporter une part de contrainte, à l'instar des mesures de police administrative qui restreignent les libertés.

Souvent condamnés à des peines sans aménagement, ces individus n'ont pas systématiquement été contraints à un suivi sociojudiciaire, la loi de 2016 n'étant pas rétroactive. Et même si certaines dispositions de la loi de juillet dernier ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020, ce dernier a lui-même ouvert la porte à un texte de remplacement en précisant, de manière très pédagogique, les motifs l'ayant conduit à juger le texte déséquilibré.

C'est tout l'objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, qui s'inscrit dans la droite ligne des dispositions antérieures. Rappelons que le Conseil constitutionnel ne s'est pas opposé au principe même de l'établissement de mesures de sûreté dans le cas de la sortie de prison des détenus terroristes, et qu'il a admis la légitimité de la mesure au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a confirmé ainsi que la mesure de sûreté n'était pas une sanction pénale dès lors qu'elle respectait un certain nombre de critères rappelés, déjà, dans sa décision du 21 février 2008. François-Noël Buffet, auteur de la présente proposition de loi, a d'ailleurs souhaité reprendre l'idée d'un suivi judiciaire postsentenciel conditionné à une évaluation de la dangerosité du condamné, et dont la durée serait fixée indépendamment de la durée des réductions de peine accordées au condamné. En définitive, c'est cet équilibre

Je le dis à cette tribune, sous le regard de Michel de L'Hospital et de Henri François d'Aguesseau, dont la rigueur n'avait d'égal que l'esprit de tolérance. C'est parce que nous veillons à l'exécution de peines proportionnées que nous mettons un point d'honneur à parfaire le droit ou à combler des carences observées. Je renverserai un célèbre adage pour vous dire ce que nous refusons tous ici en matière antiterroriste : agiter une main de velours dans un gant de fer. C'est dans cet esprit, exigeant et proactif, que nous traitons ce jour d'une problématique sécuritaire aux atours de défi civilisationnel. Je veux bien sûr saluer le travail de mes collègues Muriel Jourda et François-Noël Buffet, qui, animés par les exigences de l'État de droit, sont parvenus à corriger un vide juridique particulièrement inquiétant pour la sécurité des Français. Nous connaissons tous ici les chiffres qui nous conduisent à anticiper des sorties « sèches » qui nous inquiètent, mais nous partageons également la conviction qu'il faut aller plus loin et imaginer une réforme de structure proportionnée à un phénomène que nous ne pouvons ignorer. Je le dis à cette tribune comme représentante d'un département meurtri par l'islamisme. En effet, si nous débattons avec une telle acuité du suivi des condamnés pour terrorisme, c'est aux fins d'apporter un palliatif aux deux enjeux qui défient l'autorité de l'État et qu'il faudra tôt ou tard affronter : le sens de la peine et sa proportionnalité, d'une part ; la physionomie du milieu carcéral, physionomie du milieu carcéral, d'autre part. C'est au Sénat que nous devons l'instauration d'une peine incompressible de trente ans et la limitation drastique des conditions d'aménagement de peine. Il nous faut désormais aller beaucoup plus loin, ne serait-ce qu'au regard des nouveaux profils auxquels nous avons affaire. Le terrorisme est de plus en plus juvénile, et son traitement pénal ne peut l'ignorer. Nous savons que les crédits de réduction automatique seront supprimés si le projet de loi Dupond-Moretti est adopté en l'état. Malgré tout, c'est la question de la perpétuité réelle que nous devons aborder. Ne nous y trompons pas, en effet : incompressibilité ne rime pas avec enfermement à vie. Je rappelle que le droit interne britannique, pourtant inspiré par l',et dont personne n'oserait dire qu'il piétine les droits de la défense, ne permettait ni élargissement ni réexamen des peines de perpétuité réelle jusqu'à ce que le juge européen n'exige la clarification d'un droit pourtant souverain. Les juridictions ne doivent pas être contraintes à offrir au condamné une perspective de libération dangereuse pour la société. deuxième mal à traiter. L'instauration de cette perpétuité réelle dès le prononcé paraît d'autant plus nécessaire que la prison est marquée par une spécificité démographique notable. Selon le dernier numéro des, l'âge moyen des personnes détenues était en France d'environ 35 ans, soit 13 ans de moins que celle de la population générale. Les condamnés pour terrorisme n'échappent pas à cette réalité, bien au contraire. Il n'est que de rappeler l'âge des cinq derniers terroristes ayant frappé en France pour comprendre le défi générationnel qui est le nôtre 36, 33 et 30 ans pour ceux de Rambouillet, et Colombes, 21 ans pour l'assaillant de Nice et seulement 18 ans pour le terroriste de Conflans. Mes chers collègues, c'est aussi le « djihadisme d'atmosphère », décrit par Gilles Kepel, que nous devons aujourd'hui défier. Or, sans suivi des détenus terroristes, relais potentiels d'une idéologie qui croît souvent en prison, c'est notre jeunesse que nous exposons. Cette proposition de loi s'attaque donc courageusement aux dommages collatéraux d'un phénomène qui constitue un défi pour notre civilisation. Nous traitons aujourd'hui les conséquences d'un mal dont il faudra très vite arracher les racines. Le travail sera long, car celles-ci se propagent pernicieusement jusque dans nos prisons. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

en particulier l'intervention du garde des sceaux et de notre collègue Alain Richard, grand spécialiste du sujet. L'année dernière, j'avais soulevé le problème du suivi des terroristes sortant de prison

Si les auteurs de cet amendement peuvent souscrire de manière générale à la mise en oeuvre de mesures pour combattre ce fléau, ils émettent de très grandes réserves sur les dispositions exorbitantes du droit commun, désormais trop nombreuses, qui dépassent bien souvent leur but premier. En l'état, le renforcement des mesures de sûreté à destination des terroristes islamistes à l'issue de leur peine est trop général, tout comme l'étaient certaines dispositions de la loi SILT et antérieurement la création du Fijait qui englobe d'autres individus que les terroristes islamistes. Les auteurs de l'amendement craignent que ce régime ne s'applique aussi,, à des militants politiques- écologistes, altermondialistes, animalistes, corses, basques, etc. -, ce qui s'avérerait totalement disproportionné par rapport à l'action militante pour laquelle ils ont été condamnés.

C'est la raison pour laquelle, tout en réaffirmant leur réserve de principe à ce texte, les auteurs de l'amendement appellent à l'introduction d'une distinction entre les destructions matérielles de biens et l'atteinte volontaire à la vie humaine. Ainsi, cet amendement propose que les individus condamnés pour des atteintes aux biens soient exclus du dispositif prévu par le présent texte, conformément au principe général de proportionnalité de la peine qui prévaut en droit pénal. Quel est l'avis de la commission ? l'avis de la commission ? Je ne porterai pas de jugement sur la valeur du militantisme violent. Je voudrais simplement indiquer que, si nous adoptions cet amendement, nous ferions perdre beaucoup d'efficacité au dispositif prévu dans au dispositif prévu dans cette proposition de loi, puisque ne seraient plus concernées les infractions relatives au financement du terrorisme ou les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

envers ce que nous sommes, des citoyens libres et éclairés, la plus grande rigueur doit être de mise. La proposition de loi marque une avancée indéniable dans la reconquête de fermeté et de crédibilité. Dans cette droite ligne, cet amendement propose de compléter l'alinéa 18, en introduisant une référence explicite au niveau de risque de récidive.

En effet, il tend à préciser que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également évaluer le niveau de risque de la personne, outre sa dangerosité. Je rappelle que la mesure de sûreté ne sera applicable qu'à des personnes qui présentent une particulière dangerosité ; le texte précise que cette dernière devra être caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme. Il est par conséquent inutile de préciser de nouveau que l'évaluation de la personne devra permettre de définir le niveau de ce risque.

Cette proposition de loi expose clairement son objectif : garantir la sécurité de nos concitoyens, en permettant à la justice de mieux surveiller certains individus et d'adapter en conséquence les sanctions en fonction de l'importante dangerosité qui les caractérise. Cet amendement vise à porter à huit semaines le placement du détenu dans le service spécialisé chargé de son observation. Face aux risques indéniables de récidive de ces individus, il est impérieux de permettre aux agents de ce service de bénéficier d'un temps d'observation et d'étude

Cet amendement vise à permettre d'ordonner la mise en place de la mesure de sûreté pour une durée maximale de deux ans. Ces individus ont commis des actes visant à détruire la République, faire tomber nos institutions et assassiner lâchement nos concitoyens. Des académiques et des journalistes ont mené des enquêtes pour comprendre les phénomènes de radicalisation et de déradicalisation

Un accord a été trouvé avec l'Assemblée nationale pour fixer la durée de la mesure de sûreté à un an. Dans la mesure où le texte qui a été déposé a pour but de répondre à la censure du Conseil constitutionnel, pas de modifier l'architecture de ce qui avait été mis en place, je vous propose de retirer cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

est à Mme Esther Benbassa. Il est fondamental, pour garantir la sûreté et la sécurité des citoyens, de prévenir toute sortie sèche de détenus radicalisés. aucune mesure relative à la prévention n'est présente dans cette proposition de loi, qui contient surtout une série de mesures de sûreté dont l'utilité n'aura que peu d'effets sur le degré de radicalité de la personne au cours des prochaines années. Nous estimons qu'en matière de lutte contre la radicalisation islamiste il est important de ne pas avoir une approche fondée uniquement sur la surveillance. Le temps de la détention doit être mis à profit pour prévenir la récidive et accompagner vers la déradicalisation, voire le désengagement. Ainsi, pour faire écho au rapport sénatorial sur la radicalisation, qui a été et que j'ai eu l'honneur de corédiger avec Mme Catherine Troendlé, le groupe Écologiste -Solidarité et Territoires demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'accès aux activités de réinsertion des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste et de celles qui sont écrouées pour des faits de droit commun repérées par l'administration et les services de renseignement comme étant susceptibles de radicalisation. Quel

n'est pas très favorable à la multiplication des rapports. Il me semble que le Parlement dispose déjà de multiples moyens d'information et de contrôle de l'activité du Gouvernement.

groupe Les Républicains, la discussion de la proposition de loi tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, présentée par Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues

ni satisfaites. Ce genre de procès finit toujours par être celui de la justice. C'est la raison pour laquelle notre commission des lois a adopté un texte qui ne modifie pas le mais qui, en quelque sorte, dans le continuum de la loi Dati de 2008, va ouvrir aux victimes le droit à un procès, dans les cas où le

Il ne s'agit donc pas de juger la folie, mais de repenser, dans les rares cas où la responsabilité pénale est contestée, l'accès au juge au sens l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Nous devons trouver le moyen le plus juste d'appréhender les effets du fait fautif sur l'irresponsabilité de l'auteur d'un acte criminel ou délictuel. C'est bien au juge qu'il appartient de décider de l'irresponsabilité pénale et, singulièrement, du lien entre le fait fautif et l'irresponsabilité. Dans le prolongement de la réforme Dati de 2008, la commission des lois a donc choisi un renvoi par le juge d'instruction vers le juge du fond, à savoir le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, lorsque le fait fautif de l'auteur a causé, au moins partiellement, l'abolition temporaire de son discernement. La cause est nécessairement au moins partielle, car les causes exclusives ne se rencontrent presque jamais. L'abolition du discernement doit être temporaire, car l'abolition définitive du discernement doit continuer d'empêcher tout procès. En modifiant non pas l'article 122-1 du code pénal, mais, au contraire, le code de procédure pénale, nous apportons deux innovations majeures dans notre droit la première est la prise en compte du fait fautif antérieur sur l'abolition du discernement ; la seconde est que, dans le cas d'un fait fautif, l'abolition du discernement entraîne non pas l'irresponsabilité, mais le renvoi vers le juge du fond, qui, lui, se prononce sur l'irresponsabilité et pourra ne pas la reconnaître. On nous reproche que les tribunaux correctionnels, et, surtout, certaines cours d'assises ne prononceront pas l'irresponsabilité pénale en cas de fait fautif. Je rejette totalement cette idée qui suppose que les jurés populaires des cours d'assises seraient incapables de juger au cas par cas, ce qui est leur mission.

Cette solution, qui permettra de décider de l'application de l'article 122-1 du code pénal, est celle qui nous paraît offrir les garanties les plus importantes au regard des principes de notre droit, répondre aux interrogations légitimes de l'opinion publique et donner satisfaction aux victimes.

Par cohérence, la commission des lois a cependant choisi de prévoir que l'intoxication alcoolique ou par stupéfiant constitue un cas d'aggravation systématique des peines et délits inscrits au code pénal. On sait en effet très bien que ces intoxications sont très souvent la cause de l'irresponsabilité.

Il vous interpellera, monsieur le garde des sceaux, sur l'état de l'expertise psychiatrique, son manque de personnel et de moyens, et les difficultés des conditions d'exercice de cette mission essentielle à tous les niveaux de l'instruction et du jugement. La commission des lois La commission des lois a cherché, sur la question complexe de l'irresponsabilité, à trouver une solution équilibrée, conforme à nos principes et permettant, nous l'espérons, de progresser ensemble.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi relative à la responsabilité pénale et à l'expertise psychiatrique.

visait à modifier l'article 122-1 du code pénal ; le second, dont je suis l'auteur, prévoyait également de modifier cet article, mais visait aussi, et surtout, les conditions de l'expertise psychiatrique en matière pénale. C'est en tant qu'auteur que j'interviens donc aujourd'hui, mais- et je sais que ce n'est pas la règle habituelle dans notre assemblée -également en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Ces deux propositions de loi concernent un sujet grave : l'appréciation portée sur l'état mental d'une personne au moment des faits qu'elle est accusée d'avoir commis. d'avoir commis. Elles ont en partie été pensées en réaction à certaines affaires tragiques que nous avons encore malheureusement tous à l'esprit. Je pense ici particulièrement à l'assassinat de Sarah Halimi et à l'émotion que cet acte antisémite a suscitée dans notre pays. En tant que législateur, il nous appartient cependant d'écrire le droit non pas en réaction aux horreurs commises, mais bien pour le temps long. Concernant la rédaction de l'article 122-1 du code pénal, que l'article unique de la proposition de loi de Mme Goulet et l'article 1 de ma proposition de loi entendaient modifier, la commission des affaires sociales ne s'est pas prononcée, se montrant ouverte aux intentions exprimées par le rapporteur de la commission des lois. L'article 122-1 du code pénal pose un principe d'irresponsabilité pénale en cas d'abolition du discernement au moment des faits en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique. Il prévoit en outre le cas d'une altération du discernement. Mme Goulet souhaitait lever l'application des dispositions de cet article en cas de faute de l'auteur. Je souhaitais, pour ma part, inscrire que l'abolition du discernement ne pouvait résulter que d'un état pathologique ou d'une exposition contrainte aux effets d'une substance psychoactive. J'insiste sur la notion de « contrainte » que l'article 1 tendait à introduire. Comme plusieurs de nos collègues l'ont très justement fait remarquer en commission, il est parfois délicat, voire impossible de prévoir l'ensemble des cas possibles lorsque C'est bien au juge qu'il appartient de décider : nous devons donc faire preuve de prudence quand nous modifions les instruments du droit dont il dispose. Je constate que, sur l'initiative de son rapporteur, dont je salue le travail, la commission des lois a retenu un autre dispositif que ceux qui étaient proposés. Nous allons en discuter dans quelques minutes. J'en viens maintenant aux articles relatifs à l'expertise. Ces dispositions sont, je le rappelle, issues des conclusions des travaux menés avec notre collègue Jean-Yves Roux au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois sur l'expertise psychiatrique et psychologique. Ce rapport et les vingt préconisations qu'il formule étaient le fruit de plus d'un an de travail sur la mission peu connue des experts psychiatres ou psychologues, entre justice et santé. J'avais alors insisté sur les conditions de réalisation des expertises et les modalités d'exercice des experts, en soulignant un manque criant de moyens. Je tiens à profiter de cette tribune pour interpeller M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et le Gouvernement sur cette question. Les conditions dans lesquelles les expertises sont diligentées et réalisées ne sont parfois pas à la hauteur des enjeux que ces expertises peuvent soulever. Quant au travail des experts, force est de constater que les critères de rémunération ne correspondent pas à la complexité de certaines affaires. Je le sais, ce sujet est pour partie réglementaire et budgétaire, et il est du ressort du Gouvernement d'y travailler et d'y répondre. La proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale reprend les recommandations d'ordre législatif figurant dans ce rapport d'information. Neuf articles portent sur l'expertise ; cinq concernent l'expertise présentencielle. Nous avons ainsi souhaité concentrer l'expertise sur les seules causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale- c'est l'objet de l'article 2 -, mais aussi prévoir à l'article 3 un délai maximal de deux mois après l'incarcération pour la réalisation de la première expertise. Sur ce second sujet, je connais les réticences, mais, là encore, j'estime qu'il s'agit pour l'essentiel d'une question de moyens. Toujours en ce qui concerne l'expertise présentencielle, nous avons tenu, à l'article 4, à exclure l'expertise psychiatrique de l'examen clinique de garde à vue. Pour ce qui est des moyens des experts pour réaliser leur mission, nous avons proposé d'intégrer le dossier médical aux scellés : tel est l'objet de l'article 5. 6, nous avons souhaité mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter une contre-expertise. Les trois articles suivants ont trait à l'expertise postsentencielle. Nous avons voulu inscrire la communication systématique par le juge d'application des peines des résultats des expertises aux experts chargés de l'examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation : c'est l'objet de l'article 7. nous avons jugé nécessaire de prévoir une meilleure répartition des missions entre l'équipe chargée de l'évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité et l'expert postsentenciel. Nous avons enfin prévu la possibilité pour l'expert psychiatre postsentenciel d'assurer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération : tel est le sens de l'article 9. Enfin, le dernier article de la proposition de loi, l'article 10, vise à renforcer les obligations déontologiques des experts et prévoit une déclaration d'intérêts obligatoire. La commission des affaires sociales a adopté trois amendements qui ont également été présentés par le rapporteur de la commission des lois. Le premier, à l'article 4, tend à préserver l'obligation légale d'expertise psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles.

Pour finir, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, et en tant qu'auteur de l'une des deux propositions de loi, je tiens à souligner deux principes fondamentaux en matière de justice concernant l'état de la personne jugée. Nous devons garder à l'esprit dans ce débat que c'est bien de l'état de la personne, et de son état mental, en l'occurrence, que nous parlons. Le principe d'irresponsabilité pénale doit être regardé comme un principe fondamental de notre droit pénal. Il s'inscrit dans la tradition humaniste de notre pays et le principe selon lequel « on ne juge pas les fous Enfin, je rappelle que le droit à un procès équitable est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et que nous devons toujours avoir à l'esprit

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, la décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021, qui a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Sarah Halimi-Attal, n'a pas été comprise. Elle a suscité une très forte et très légitime émotion.

D'une part, l'abolition du discernement de l'auteur d'un homicide peut aujourd'hui résulter de son intoxication volontaire, notamment après l'absorption de substances stupéfiantes.

que les dispositions de l'article 122-1, premier alinéa, du code pénal ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement ». Je voudrais d'ailleurs me joindre à votre hommage,

dans cette enceinte, lors d'un débat organisé sur l'initiative de votre groupe, madame la rapporteure, il était nécessaire d'attendre l'énoncé de la Cour de cassation. Celle-ci a désormais dit les choses clairement : le juge ne peut distinguer là où le législateur ne le fait pas. Comme je l'ai annoncé voilà quelques semaines, j'ai mené à la suite de la prise de parole du Président de la République une large consultation sur la modification du régime de l'irresponsabilité pénale. J'ai reçu les représentants des cultes, des magistrats, des experts psychiatres, des professeurs de droit. Il s'agit d'un sujet éminemment complexe et vous-même, madame la rapporteure, avez pu évoluer dans votre appréhension de la réponse à apporter, dans un sens que, d'ailleurs, de ces consultations, et des avis concordants qui en sont issus, je vous rejoins sur le fait que l'article 122-1 du code pénal ne doit pas être modifié. Article fondamental de notre droit positif, il est et doit rester le garant du principe essentiel posé par l'article 121-3 du même code : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » Dans notre pays, comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom, on ne juge pas les fous. Revenir sur ce principe serait une régression insupportable, une ligne rouge qui ne doit pas être franchie Cette cause traditionnelle d'irresponsabilité pénale répond à une exigence juridique, constitutionnelle et conventionnelle, qui est essentielle dans tout État de droit respectueux des libertés individuelles et de la personne humaine, et qu'il n'est nullement question de remettre en cause. Je le dis et le redis, il n'est pas envisageable de condamner une personne pour un acte commis alors qu'elle ne disposait pas de son libre arbitre. Nos débats nous permettront néanmoins d'échanger sur le contenu de l'article 1 de la proposition de loi, tendant à prévoir l'organisation systématique d'un débat devant la juridiction de jugement lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en cause résulte au moins partiellement de son fait fautif. Mais, du fait de la sensibilité toute particulière du sujet qui nous réunit aujourd'hui, il me semble indispensable de bénéficier des éclairages du Conseil d'État. J'ai donc souhaité disposer de son avis éclairé avant toute modification éventuelle du régime d'irresponsabilité pénale. C'est pourquoi, comme je m'y étais engagé, le Gouvernement vient de soumettre à l'examen de celui-ci un projet de loi qui permettra de limiter l'irresponsabilité pénale lorsque l'abolition du discernement résulte d'une intoxication volontaire. les sénateurs, que dans l'attente de cet avis du Conseil d'État, je me borne aujourd'hui aux quelques observations suivantes sur le texte proposé par votre commission. Je tiens d'abord à saluer l'important travail réalisé par ses soins et les modifications apportées au projet initial. Nous nous rejoignons désormais sur la nécessité de ne pas modifier les règles posées par l'article 122-1 du code pénal et de maintenir l'irresponsabilité pénale en cas de disparition du libre arbitre. Mais pourquoi, comme prévu dans la proposition de loi, saisir la juridiction de jugement, notamment la cour d'assises ? Est-ce pour permettre aux jurés d'écarter l'article 122-1, car ils estimeraient que le discernement de la personne était simplement altéré, et non aboli ? ? Si les experts et le juge d'instruction ont conclu à l'absence de doute sur l'abolition du discernement, ce renvoi ne me semble pas justifié. Est-ce pour permettre aux jurés de considérer que les dispositions de l'article 122-1 ne devraient pas s'appliquer, au motif que la disparition du libre arbitre résulte d'une consommation illicite, et donc fautive, de stupéfiants ? Il faudrait alors que cette exception soit explicitement prévue par la loi ! Je suis par ailleurs très réservé sur les dispositions de l'article 2 de cette proposition de loi, tendant à insérer une disposition générale d'aggravation des peines en cas d'infraction commise « en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants ». Cette aggravation existe déjà dans de nombreux cas, comme les violences, le viol ou les agressions sexuelles. Elle pourrait sans doute être prévue pour d'autres infractions comme le meurtre. Mais la généralisation souhaitée ne va-t-elle pas à l'encontre de l'objectif visé, en banalisant pour toutes les infractions,

Après analyse, certaines ne me semblent pas relever de la loi et peuvent susciter des interrogations. S'il est évident qu'une expertise psychiatrique doit intervenir aussi rapidement que possible,

L'impossibilité de procéder, hors délai, à cette expertise ? Et si la personne n'est arrêtée que plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, ce délai de deux mois a-t-il encore un sens ? encore un sens ? J'en viens à l'article 10 et aux obligations déontologiques des experts. Je tiens à préciser que celles-ci rejoignent pleinement les projets d'amélioration sur lesquels j'ai demandé aux services de la Chancellerie de travailler. Il importe effectivement d'éviter des conflits d'intérêts lorsqu'une personne est chargée d'une expertise, et cette question dépasse évidemment la seule hypothèse des expertises psychiatriques. L'expert doit donc faire connaître ses activités professionnelles ou bénévoles, ainsi que ses fonctions ou mandats électifs, passés ou en cours, susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Mais il ne me semble pas pertinent, comme proposé à l'article 10, d'imposer à l'expert des déclarations avant chacune de ses expertises, pas plus qu'on ne demande une déclaration d'intérêts aux magistrats avant chaque décision, ou aux parlementaires avant chaque vote. Mesdames, messieurs les sénateurs, comme pour le texte précédent sur les sortants de prison, j'observe que nous travaillons sur des projets parallèles et, en réalité, très complémentaires. J'y vois un nouveau témoignage de l'implication conjointe du Sénat et du Gouvernement sur les sujets d'importance pour nos concitoyens. Je rappelle, pour être complet, que la commission des lois de l'Assemblée nationale a lancé de son côté une mission « flash sur le sujet de l'irresponsabilité pénale. L'occasion m'est donc à nouveau donnée de saluer la mobilisation des deux chambres du Parlement. Toutefois, le travail engagé par le Gouvernement sur la question de l'irresponsabilité pénale, désormais soumis à l'avis du Conseil d'État, me semble mieux à même de répondre à la problématique posée par la décision de la Cour de cassation.

Je n'en doute pas, les propositions concrètes formulées aujourd'hui par le Sénat viendront utilement nourrir le projet de loi qui vous sera présenté prochainement.

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, certains nous reprocheront de légiférer sous le coup de l'émotion et d'autres salueront la volonté du législateur de se saisir de sujets complexes mis en avant par l'actualité. Sans nier l'émotion de ces derniers mois suscitée l'affaire Sarah Halimi, je regrette que notre chambre n'ait su éviter certains écueils dans le travail accompli sur la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui. Certes, le sujet et son traitement sont délicats. Le questionnement au coeur des débats est bien celui de la prise en compte, ou non, du fait fautif entraînant l'abolition du discernement, bien sûr sous-tendue par l'envie, le besoin même des victimes de voir l'affaire jugée publiquement. L'article 1 de la présente proposition de loi tente de répondre du mieux possible, mais, me semble-t-il, de manière incomplète, à cette problématique. Il introduit la recherche du fait fautif dans l'abolition du discernement, mais seulement au niveau du code de procédure pénale, dans le seul but de renvoyer au juge du fond la tâche de déclarer, ou non, le mis en cause responsable pénalement. Si le but était d'enjoindre le juge à exclure l'irresponsabilité pénale en cas de fait fautif,

Venons-en au besoin d'un procès, que nous devons prendre en considération. L'audience en chambre de l'instruction, qui se concentre sur la question de la responsabilité pénale du mis en cause, est déjà publique et contradictoire, en présence des victimes et avocats des parties civiles. Collégialité de la décision et possibilité d'expertise créent une configuration qui paraît respectueuse de notre système pénal. Nous devons toutefois, en tant que législateur, rester d'une extrême vigilance pour manier et différencier les notions et les règles d'imputabilité et de responsabilité. Clairement, la notion que le doute doit bénéficier au mis en cause est fondamentale dans notre système pénal, mais ne peut s'appliquer qu'à l'accomplissement même des faits, donc à l'imputabilité. La question de la responsabilité pénale atténuée, abolie, ou pleine et entière, est d'une tout autre nature. Loin de nier qu'il existe des degrés entre la responsabilité et l'irresponsabilité, comment juger ? C'est à l'aune de cette capacité d'en juger que se pose la question du fait fautif antérieur. Oserons-nous cheminer, sur le plan philosophique et technique, vers ce que certains appelleraient le concept de « folie volontaire » Certes, un comportement volontaire peut directement contribuer au déclenchement de l'abolition du discernement, mais ce trouble fort a-t-il été envisagé ou souhaité ? Le juge, faisant appel aux expertises psychiatriques, est celui qui jugera de l'engagement de la responsabilité et de son atténuation. Ne compliquons pas son magistère en lui imposant de renvoyer au juge du fond, dès qu'il y a un fait fautif- je dirais même : dès qu'il « estime » qu'il y a un fait fautif. Cette responsabilité du mis en cause devient bien trop complexe. Il connaîtrait précisément le risque et l'aurait volontairement pris dans un dessein criminel ... Comment, réellement, scientifiquement, sûrement, connaître les risques et conséquences d'une toxicologie qui est différente selon les personnes, les moments, les associations de substances ? Qui, ici, pourrait affirmer qu'il est toujours possible de constater et d'évaluer la part de la cause endogène ou exogène du trouble ayant conduit à l'abolition du discernement ? Cette ligne de crête

loi vise, lui, à augmenter les peines pour les crimes et délits commis en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants. Là encore, j'entends l'idée de punir plus sévèrement ce que nous pouvons percevoir comme un fait fautif : l'absorption de stupéfiants ou d'alcool. C'est déjà, souvent, ce que font les juges- on estime que, pour la moitié des faits de violences conjugales, l'alcool ou les stupéfiants sont impliqués. Mais je reste prudent sur ce point, redoutant une tendance à privilégier de plus en plus la pénalisation des addictions sur une prise en compte plus globale en termes de santé publique. Je salue, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, l'ensemble des autres articles qui s'attachent au problème récurrent de notre système judiciaire : il nous faut donner de vrais moyens pour les expertises psychiatriques. De la lenteur pour effectuer les expertises aux dysfonctionnements des barèmes de paiement, à la facilitation du secret médical partagé : il était urgent d'agir. Le temps passe et je souhaite conclure en appelant notre assemblée à une très grande prudence : nous nous devons de prendre du recul sur l'émotion, justifiée, de l'opinion publique. Nous devons préserver la notion d'irresponsabilité pénale, même si celle-ci devient de plus en plus insupportable pour la population, acceptant mal que certaines personnes ne puissent être jugées et condamnées pénalement pour leurs crimes. Pour autant, le mis en cause passe devant la justice et il est soumis aux décisions des juges, notamment l'hospitalisation sous contrainte. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne votera pas ce texte.

le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des travaux du Sénat sur le sujet complexe et important de l'irresponsabilité pénale, un sujet à la frontière du monde juridique et du

Je pense aussi à la mission d'information pluraliste de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, dont notre rapporteur pour avis était l'un des rapporteurs, qui s'est en grande partie concentrée sur l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Elle a formulé, en mars dernier, des propositions intéressantes afin d'améliorer les conditions de réalisation de l'expertise, ainsi que sur la déontologie des experts. C'est donc dans une certaine continuité et avec cohérence que le Sénat se saisit aujourd'hui de la question de l'irresponsabilité pénale au travers de deux points : son régime, d'une part, et l'expertise psychiatrique qui s'y rattache, d'autre part. Cette continuité ne saurait, bien sûr, s'abstraire des décisions rendues à la suite du meurtre, d'une violence saisissante et inacceptable, de notre concitoyenne Mme Attal-Halimi. Notre détermination doit être totale pour lutter contre les surgissements de l'antisémitisme, dont Mme Attal-Halimi a été la victime,

Il nous faut réfléchir au dispositif le mieux à même de persévérer dans notre État de droit juste, fraternel et protecteur. Nous nous trouvons à l'intersection d'impératifs distincts, d'égale importance et parfois difficilement conciliables

Sur le fondement de cette recherche d'équilibre, notre assemblée, tout comme le Gouvernement, a réaffirmé son intention d'apporter une réponse à l'étonnement légitime face aux situations auxquelles le droit en vigueur peut conduire. Ce cheminement n'est pas un tâtonnement, tiède ou feint ; il est la marque d'un travail approfondi et nécessaire au regard de l'enjeu. La dernière grande réforme, qui permet à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la matérialité des faits à l'issue d'un débat public et contradictoire, y compris lorsque ceux-ci s'appuient sur des représentations de haine telles que l'antisémitisme, tout en retenant l'irresponsabilité pénale de leur auteur, montre bien toute la complexité du régime de l'irresponsabilité et des actions entreprises pour le faire évoluer. À ce titre, le choix de nos rapporteurs de ne pas conserver la révision de l'article 122-1 du code pénal initialement envisagée- dans une rédaction d'ailleurs différente de celle que proposait, un mois plus tôt, la mission d'information du Sénat -s'entend. Désormais, l'article 1 prévoit donc que, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement résulte au moins partiellement du fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement, qui statuera sur l'irresponsabilité pénale et, le cas échéant, sur la culpabilité. Des interrogations ont pu être exprimées en commission sur la portée de cette réécriture. Il faut rappeler que la compétence des juges du fond pour statuer sur l'irresponsabilité de l'auteur des faits, notamment la compétence des cours d'assises et de leur jury, est déjà prévue par le droit en vigueur dans le cas où les juges d'instruction ont considéré que l'auteur était responsable pénalement. L'article 1 viserait donc à faire intervenir la juridiction de jugement en amont, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte au moins partiellement de son fait fautif. L'objet serait ainsi de garantir un « vrai procès aux victimes », pour reprendre les mots de Mme la rapporteure, tout en ne renvoyant devant la juridiction de jugement que les personnes en état de comparaître. Deux points peuvent être relevés, avec toute la prudence que la complexité du sujet implique. D'une part, peut-on continuer de se poser la question de l'appréciation du fait fautif par la chambre de l'instruction ? C'est une question importante, car la portée du dispositif en dépend. S'il est difficilement compréhensible pour la société qu'une personne puisse être exonérée de sa responsabilité pour un état résultant d'une attitude délibérée, comment qualifier l'addiction ? Est-elle une faute ou devient-elle, dans la durée qui lui est inhérente, une contrainte subie ? Le sujet est d'autant plus délicat qu'il déborde la matière pénale et intègre à la réflexion les politiques de santé publique et de prévention. envisager d'autres voies pour répondre au besoin des victimes d'avoir un « vrai procès ». Je pense, par exemple, à une modification des modalités de l'audience publique devant la chambre de l'instruction, instituée en 2008, pour en renforcer le caractère contradictoire. Houillon et Dominique Raimbourg sur l'irresponsabilité pénale a d'ailleurs préconisé plusieurs ajustements de cette réforme. Une autre difficulté réside dans le placement du curseur entre l'abolition et l'altération du discernement, notion finalement assez récente dans le régime de l'irresponsabilité puisqu'elle a été introduite en 1994 seulement. En tout état de cause, le choix de Mme la rapporteure d'entrer par la voie d'une révision de la procédure contribuera au cheminement entrepris pour aboutir à une solution dont les différentes parties entendent aujourd'hui la nécessité.

Elle n'est pas revenue sur la décision de la cour d'appel de Paris, marquant certes une continuité jurisprudentielle, mais suscitant une colère, une indignation et des interrogations qu'il est aisé de comprendre. Toutefois, la lecture de cet arrêt est riche d'enseignements, car elle met au jour deux thèses radicalement opposées. D'un côté, la thèse retenue par les juges, appuyée sur les expertises psychiatriques et appliquant la mécanique de la responsabilité pénale, conclut à l'irresponsabilité pénale de M. Kobili Traoré. Ainsi, au regard de la vérité judiciaire, ce dernier demeurera sujet à des bouffées délirantes. À ce titre, l'arrêt précise : « [ ...] Aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation. De l'autre côté, la thèse des auteurs du pourvoi, la famille de Sarah Halimi, fait valoir que le seul fait de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience de leurs effets potentiels sur le discernement, devrait exclure la prise en considération de l'abolition du discernement. À l'inverse, l'acte volontaire de consommation de stupéfiants devrait être constitutif d'un comportement fautif excluant l'irresponsabilité. Cette seconde solution est bien sûr compréhensible ; est-elle trop radicale pour qu'un juge la retienne ? Sans doute. Si l'on ne peut laisser à une juridiction la responsabilité d'un tel revirement, c'est au législateur de se pencher Il revient donc au Parlement de déterminer comment exclure du champ d'application de l'irresponsabilité pénale les cas dans lesquels la faute de l'auteur est à l'origine de son état d'irresponsabilité. La proposition de loi élaborée par notre collègue rapporteur Nathalie Goulet et celle cosignée par nos collègues membres des commissions des lois et des affaires sociales inaugurent cette réflexion. Je me réjouis que le Sénat soit à l'initiative de ce travail. Les premiers échanges auxquels il a donné lieu en révèlent toute la complexité. La solution la plus instinctive serait de modifier l'article 122-1 du code pénal, qui édicte le principe de l'irresponsabilité pénale d'une personne personne atteinte, « au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Seulement, l'article 122-1 pose un

De ce point de vue, je tiens à saluer le travail effectué par la commission des lois : cette dernière a retenu une solution alternative plus respectueuse de nos principes. La procédure proposée pourrait effectivement permettre d'éviter certaines incompréhensions, dans des cas aussi dramatiques que le meurtre de Sarah Halimi.

rendu par nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux à la suite des auditions menées par un groupe de travail dont j'approuve entièrement l'initiative. En effet, ce groupe de travail a été constitué lors de la précédente mandature, à ma demande, alors que j'étais membre du bureau de la commission des lois, et avec l'appui de son président d'alors, Philippe Bas. Aussi, je remercie sincèrement Jean Sol de m'avoir associée à la signature de la proposition de loi issue de ses travaux, qui étaient très attendus. Cette proposition de loi reprend près de la moitié des préconisations que nous avons formulées et que je cite pêle-mêle lever les blocages dans la communication des dossiers médicaux ; mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise ; renforcer l'information des experts ; ou encore renforcer les obligations déontologiques de ces Ces évolutions sont vivement espérées. Nous saluons donc l'ensemble des propositions retenues : au regard de ces dernières, le groupe RDSE, très impliqué dans ces questions, se prononcera avec force et conviction pour le présent

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, des affaires tragiques- le meurtre de Mohamed El Makouli en janvier 2015 et, plus récemment, celui de Sarah Halimi le 3 avril 2017

pénale. Dans les deux cas, les avocats des parties civiles ont invoqué la prise antérieure de stupéfiants pour contester l'abolition du discernement au moment des faits et donc l'irresponsabilité pénale. En application de l'article 122-1 du code pénal, cette détermination relève de l'appréciation souveraine des juges. Toutefois, celle-ci est contestée sur un point précis la prise en compte du fait fautif de l'auteur de l'acte, autrement dit la consommation de stupéfiants ou d'alcool antérieurement à la commission de l'infraction. En la matière, la jurisprudence est constante. Elle montre que ce fait fautif n'a jamais été reconnu, puisque l'intention de l'auteur s'apprécie au moment des faits. Mais il s'agit là d'un vieux sujet de controverses en doctrine et, surtout, dans l'opinion publique. C'est dans ce contexte que la commission des lois a souhaité mettre à l'ordre du jour la question de l'irresponsabilité pénale en examinant deux propositions de loi en une.

Je pense notamment à l'article 4, qui restreint le champ de l'examen clinique prévu en garde à vue à la compatibilité de santé de la personne avec la mesure. En revanche, nous sommes vertement opposés au principal dispositif proposé. nous pouvons nous réjouir que l'article 122-1 du code pénal reste finalement intact, comme le préconisait d'ailleurs le rapport de MM. Raimbourg et Houillon. Mais la rapporteure n'a pas abandonné l'idée selon laquelle, lorsque l'auteur d'un crime ou d'un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l'abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue. Ce mécanisme emporte deux conséquences non négligeables et même, selon nous, déplorables. Premièrement, il vise à instaurer, dans certains cas, un véritable procès d'abolition du discernement, alors même qu'une audience publique est prévue par la loi de 2008. À nos yeux, ce procès symbolise le rapport disciplinaire entre justice et folie. Pis, il exhiberait la souffrance de toutes les parties sans permettre la « consolation parfois espérée. D'ailleurs, on peut déjà le constater lors des audiences publiques. Aussi, je m'interroge : cette forme de procès pour les personnes qui relèvent de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne ferait-elle pas fléchir l'institution vers une justice que je qualifierai d'outrancière ? malgré les précautions prises avec la notion d'abolition temporaire, les garanties du procès équitable, qu'exige notamment le droit international, ne sont pas observées. Deuxièmement, avec ce mécanisme de fait fautif, l'irresponsabilité pénale ne sera plus automatique lorsqu'on sera face à une abolition du discernement. S'ajoute donc, aux notions d'altération du discernement et d'abolition, la notion d'abolition temporaire liée à un fait fautif. Légiférer en ce sens, ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs

Mais la responsabilité du politique, c'est-à-dire de nous tous ici présents, ne serait-elle pas de dépassionner le débat judiciaire, de mettre en place des pare-feux juridiques pour protéger les plus faibles au lieu d'alimenter ce débat judiciaire de commentaires politiques opportunistes, voire de propositions de loi de circonstance ? Pourtant, contrairement au soin, la peine a une fin. L'univers d'une unité pour malades difficiles est aussi privatif de liberté que l'univers carcéral. L'unique différence est que le personnel qui y exerce est Finalement, à l'heure où l'équilibre entre sécurité et liberté n'a jamais été aussi fragile, nous voyons à l'oeuvre un courant d'utilitarisme pénal qui se mue, depuis des années, en populisme pénal. Ce texte en est l'énième illustration, bien que que les doutes profonds exprimés par la commission des lois et l'ensemble des juristes qui y siègent soient le reflet de la difficulté majeure à surmonter en la matière : depuis le droit romain et le Talmud, « on ne juge pas

intérêt, cette proposition de loi dans son économie générale traduit une vision de la société qui n'est pas la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous la rejetterons

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues,

que son auteur est irresponsable. En résulte une question que chacun se pose : comment un acte irresponsable peut-il être antisémite ?

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

en présence des parties et de l'auteur du crime, et en plein respect du contradictoire. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a pas eu de procès.

la juridiction de jugement statuerait sur la question de la responsabilité avant l'examen au fond.

aux fins de commettre l'infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. » Tout en maintenant

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a de grands principes qui fondent notre droit et qui se confrontent : on ne soumet pas à un procès les individus n'étant pas en capacité de présenter personnellement leur défense ; on ne juge pas les fous. Cependant, on a le devoir de mettre hors d'état de nuire les individus dangereux et celui d'assurer aux parties civiles que justice soit faite quand le mal est fait. L'irresponsabilité pénale ne doit être invoquée qu'en cas d'extrême nécessité, car la justice et la sécurité doivent être assurées. Mais depuis dix ans le nombre d'ordonnances d'irresponsabilité a fortement augmenté. Ce terme et, surtout, sa signification ne doivent pas être dévoyés. Or il semble que la culture de l'excuse soit aussi florissante que la culture du cannabis. Je pense tout spécialement à la douleur de la famille de Sarah Halimi le 14 avril dernier, jour où les juges de la Cour de cassation ont confirmé que le meurtrier était pénalement irresponsable au moment des faits ; qu'il était en proie à une « bouffée délirante » lorsqu'il a tué sa voisine, après la consommation de stupéfiants. Ce criminel ne sera pas jugé, car les juges ont estimé que fumer du cannabis en quantité et tuer une personne juive aux cris d'« Allah Akbar n'était que la « bouffée délirante » passagère d'une personne tout à fait normale, refusant de voir qu'il était activement en proie à des bouffées islamistes, antisémites et criminelles. Résultat : ni prison ni hôpital psychiatrique pour Kobili Traoré ; une bouffée de haine de plus dans la nature. Que se passera-t-il s'il récidive ? Il y a la séparation des pouvoirs, mais nous sommes là aussi pour exprimer la colère d'une famille et de la famille nationale, pour faire en sorte que le code pénal et le code de procédure pénale ne légitiment pas la culture de l'excuse. Abolir volontairement son discernement par la consommation volontaire de drogues, n'est-ce pas déjà avoir fauté ? ? La tolérance croissante de notre société face aux substances psychoactives et aux drogues nous expose à ces excès, à ces drames et à ces injustices. Alors que le débat sur la légalisation du cannabis s'est invité au Parlement, au point que l'on a pu voir un député brandir un joint dans l'hémicycle à croire qu'il venait d'en fumer un ... -, les parlementaires doivent considérer l'expression de la responsabilité dans le droit en questionnant d'abord leur propre qualité de responsable politique. Au-delà des évolutions législatives, il est bon que le sentiment d'injustice né de l'absence de procès et de jugement se fasse entendre par l'institution judiciaire elle-même : car c'est elle qui voit, entend, touche et doit comprendre le pays réel. Il convient ensuite de donner aux juges, dans leur appréciation souveraine, les moyens financiers et humains nécessaires pour rendre la justice et mieux éclairer leur jugement. Il y a une dernière condition pour que la justice soit rendue : son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, qui plus est lorsque le ministre de tutelle se vante d'être le ministre des délinquants

comme nous tous, j'ai une pensée émue pour Sarah Halimi et les membres de sa famille. Son meurtre est une tragédie. La proposition de loi que nous examinons dépasse le cadre de cette affaire : pourtant, c'est bien ce meurtre qui a mis l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au centre de l'actualité. Mal comprise, l'irresponsabilité pénale choque parfois. Certains y voient une forme d'immunité, voire une incitation au crime. Or la réalité est bien différente. Il faut admettre que les troubles psychiques, même dangereux, ne se traitent pas avec une sanction pénale. La place de ceux qui en sont atteints est à l'hôpital et non pas en prison. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent être remis en liberté. Quand le meurtrier de Mme Halimi a été déclaré irresponsable, la juridiction juridiction a « ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté ». L'objectif principal des auteurs de cette proposition de loi était de restreindre le champ d'application de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Nos collègues souhaitaient empêcher que puissent être déclarés irresponsables ceux dont le comportement est à l'origine du trouble mental. Leur initiative s'inscrit dans le sillage d'autres réflexions. Un projet de loi sur la question sera prochainement présenté et une mission flash est en cours sur le sujet à l'Assemblée nationale- les précédents orateurs l'ont déjà rappelé. Le travail en commission, notamment les auditions menées dans le cadre de l'examen du présent texte, a montré toute la difficulté qu'il y a à tenter de rendre quelqu'un responsable de son irresponsabilité. Nos collègues n'ont eu d'autre choix que de renoncer à modifier la règle de l'irresponsabilité pénale : aucune rédaction ne permettait d'éviter une atteinte aux principes fondamentaux de notre droit. je salue la décision de la commission. C'est une décision de sagesse, qui ne laisse pas l'émotion, même légitime, prendre le pas sur l'intérêt général. Avec sa rédaction, la commission nous propose d'améliorer plusieurs points de procédure du domaine de l'expertise judiciaire. Ces améliorations sont les bienvenues. Celle qui permet d'écarter tout conflit d'intérêts de la part de l'expert nous semble particulièrement pertinente. En outre, le texte de la commission contient une disposition visant à ce qu'un procès pénal se tienne lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte de son fait fautif. La responsabilité pénale serait déterminée lors de ce procès afin de faire droit au besoin de procès des victimes. Bien entendu, l'objectif est louable et nous tenons à ce que la place des victimes soit respectée. Toutefois, nous craignons que cette solution n'entraîne encore davantage de frustration : tenir un procès pour finalement déclarer l'auteur irresponsable ne sera pas plus facile pour la partie civile. Par ailleurs, il semblerait que des doutes persistent quant à la solidité juridique de la rédaction proposée. Cette disposition nous inspire donc quelques réserves. Enfin, le texte entend préciser pour l'ensemble des infractions que la consommation d'alcool ou de stupéfiants est une circonstance aggravante.

n'était pas prévue pour certains crimes pourtant particulièrement graves, comme la torture et les actes de barbarie. Il nous paraît indispensable de l'étendre à l'ensemble des crimes et délits. et délits. Ainsi, le message sera clair : la consommation d'alcool ou de stupéfiants, loin d'excuser le comportement de l'auteur, renforce la peine qu'il encourt. ce texte contribue à l'amélioration de notre droit pénal. Si nous ne souscrivons pas à l'ensemble de ses mesures, nous sommes particulièrement favorables à un renforcement des sanctions à l'encontre de ceux qui commettent des infractions sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool. Nous soutiendrons donc l'adoption

le meurtre de Sarah Halimi nous a tous choqués. Nombreux, nous attendions le procès de son meurtrier pour mieux comprendre comment s'est développé et comment se développe encore cet antisémitisme qui touche certains de nos jeunes mieux le comprendre pour mieux le combattre, en donnant un signal fort grâce à un vrai procès. Le racisme n'a pas de raison d'être, l'antisémitisme n'a pas de fondement et nous nous de lutter contre ces fléaux afin de préserver notre unité et de faire Nation. Nous attendions ce procès pour montrer que la bêtise peut se transformer en haine, la haine en violence meurtrière, et que la violence est punie par la loi. Nous attendions ce procès pour dire la justice : la justice pour Sarah, la justice pour sa famille, la justice pour nous tous. Or, de procès, il n'y a pas eu ; enfin, pas un vrai procès d'assises avec des jurés, en présence de l'accusé. Le meurtrier, en plus d'être antisémite, était drogué et c'est bien la somme de tout cela qui l'a conduit à tuer Sarah Halimi. Mais, au moment des faits, une bouffée délirante lui a ôté son discernement et si l'on peut juger les imbéciles, les méchants et les violents, on ne juge pas les fous. Aucun des experts qui se sont prononcés dans cette affaire n'a remis en question la folie du meurtrier au moment de son crime. Mais aucun des experts n'a mis en doute le fait que le cannabis à haute dose consommé par le meurtrier y était pour quelque chose. La seule question était : une maladie mentale a-t-elle été exacerbée par la drogue ou est-ce la drogue qui a conduit à la maladie mentale ? Il s'agit là d'un débat la justice, une seule chose à retenir : le meurtrier n'avait plus de discernement au moment des faits, celui-ci ayant été aboli par sa consommation volontaire de cannabis, c'est-à-dire de son propre fait, en l'occurrence fautif. Nous voici donc au point qui nous préoccupe. L'article 122-1 du code pénal, qui permet de déclarer un auteur pénalement irresponsable, devait-il s'appliquer à une personne dont le discernement a été altéré de son propre fait ? Que ce soit de son fait ou non, l'auteur était irresponsable au moment du meurtre et cela, nous ne pouvons rien y faire. Devrait-on le juger pour des faits qu'il n'a pas commis en toute conscience ? Jusqu'à présent, notre droit et notre justice s'y sont toujours refusés, malgré les propositions faites en ce sens par certains spécialistes. Notre rapporteur nous propose de rester sur cette ligne. Malgré l'émoi suscité, nous nous devons de légiférer avec le recul nécessaire, en laissant de côté notre émotion légitime. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions et, en particulier, de nous demander si l'approche mise en oeuvre ne devrait pas être différenciée entre un auteur rendu meurtrier par sa propre faute et un auteur que le libre arbitre a quitté sans qu'il ait rien fait pour. Le premier ne pouvait ignorer que son comportement pouvait le pousser à ne plus se maîtriser ; le second est une victime collatérale de son propre état.

On sait que la justice est réparatrice pour les victimes, même si, dans le cas présent, elle ne ramènera pas une mère. Le fait que la culpabilité de l'auteur soit reconnue permet de conférer aux personnes qui ont subi ses actes le statut de victime ; c'est pour cela que le jugement est l'objet de cette proposition de loi. Il s'agit de permettre que le jugement ne se limite pas à la décision de la chambre de l'instruction, comme c'est le cas en l'espèce, ou à l'ordonnance du juge d'instruction, mais que, lorsque l'auteur est à l'origine de l'abolition de son propre discernement, on rende tout de même justice aux victimes par un procès public. Dans le cas Halimi, que se serait-il passé ? Un procès public aurait eu lieu, durant lequel l'auteur aurait, comme il l'a fait devant la chambre de l'instruction, reconnu son crime et présenté ses excuses aux victimes. Il aurait, très probablement, été déclaré irresponsable de la même façon. Les victimes, elles, auraient été reconnues publiquement et la cour aurait pu rappeler, également publiquement, avec un écho plus large que celui de la chambre de l'instruction, que l'antisémitisme est pénalement répréhensible. Pour la suite, l'auteur est en hôpital psychiatrique et sa seule sanction est de ne plus apparaître dans le périmètre géographique de son crime pendant vingt ans. Pourrait-il sortir libre dès demain, sans obligation de soins, sans être contraint de ne jamais retoucher à une quelconque drogue ? qui devront y répondre, alors que, à mon sens, le juge devrait pouvoir intervenir à ce moment, afin de prendre en compte la dangerosité potentielle de la personne que l'on aura à libérer un jour, si elle va mieux. On ne juge pas les fous, c'est juste, mais savoir mesurer leur dangerosité et s'en protéger, c'est également justice. Notre groupe salue l'initiative de nos deux collègues Nathalie Goulet et Jean Sol, qui nous donne l'occasion d'avoir aujourd'hui un débat nécessaire sur l'évolution de l'irresponsabilité pénale, mais également sur ce qui permet de la caractériser : l'expertise psychiatrique du prévenu ou de l'accusé. Grâce à leurs travaux, nous aboutissons aujourd'hui à un texte équilibré que notre groupe soutiendra,

en tant que législateur, il est des combats que nous pouvons mener, des réponses que nous pouvons apporter, des besoins que nous pouvons satisfaire ; il en est d'autres pour lesquels la réponse est plus malaisée. La question de l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques exige ainsi beaucoup d'humilité.

En sympathie avec les proches des victimes, nous percevons le caractère incommensurable de leur douleur ; nous partageons leur besoin de comprendre, leur soif de justice, leur volonté d'obtenir réparation. Comme les leurs, nos questionnements et nos exigences restent insatisfaits, car, si la justice commande qu'un auteur réponde de ses actes devant la société, l'irresponsable, au sens étymologique du terme, n'en a pas la capacité et laisse la société, comme les victimes, sans réponse. réponse. Je n'oublierai ainsi jamais, parce que cela s'est passé sur le territoire de la commune dont j'étais le maire, ces deux familles détruites après qu'un jeune homme atteint de schizophrénie a tué sa petite amie. L'irresponsabilité n'efface pas l'horreur du crime, elle y ajoute l'incompréhension face au « crime du fou ». Ces histoires dramatiques nourrissent une insatisfaction profonde et un débat public sur ce qui pourrait changer. Or la voie est étroite et l'on peut envisager les choses d'un tout autre point de vue. Ainsi que l'a rappelé Jean Sol, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, les travaux communs de nos deux commissions étaient, à l'origine, d'une autre nature. Il s'agissait, à la demande de notre collègue Nathalie Delattre, d'examiner les conditions de l'expertise psychiatrique en matière pénale sur la base du constat que la santé mentale de nombreuses personnes incarcérées est défaillante, que ces dernières aient été atteintes de troubles mentaux avant leur procès ou qu'elles en aient développé par la suite. L'angle de départ était plutôt que ces malades mentaux n'avaient pas forcément leur place en prison. Au-delà de la misère de la psychiatrie en France, déjà bien documentée par de nombreuses analyses, les travaux de nos commissions ont mis en lumière les grandes difficultés de l'expertise psychiatrique, s'appuie sur une ressource de plus en plus rare, et néanmoins plutôt peu et mal pilotée. C'est ce à quoi l'essentiel de la proposition de loi de Jean Sol s'efforçait de remédier. Je ne voudrais pas, monsieur le garde des sceaux, que le débat sur l'irresponsabilité pénale occulte totalement cette partie du texte. Dans cette matière, certes moins noble et plus concrète, il est évident que le ministère de la justice doit progresser. Nous partons de loin : la commission a, par exemple, réalisé, il y a peu, que le dossier du travail des experts ne semblait tout simplement pas géré par la Chancellerie.

Avec Jean Sol, nous avons considéré que la question de l'intoxication volontaire par des substances psychoactives devait être posée. L'irresponsabilité ne doit pouvoir être retenue que lorsqu'elle n'a pas été expressément recherchée. C'est pourquoi la rédaction proposée dans la proposition de loi retenait la notion « d'exposition contrainte aux substances psychoactives », seule susceptible d'entraîner une abolition du discernement. rédaction préservait également la capacité du juge à apprécier les circonstances de l'espèce, ce qui me semble indispensable, le législateur ne pouvant tout prévoir, énumérer tous les cas de figure dans la loi et encore moins se substituer au juge ou à l'expert, même si, sous le coup de l'émotion, il peut en éprouver le besoin. Il est, en revanche, une responsabilité qu'il porte, celle de créer les conditions d'une prise en charge correcte de la santé mentale dans notre pays et, même si je connais moins bien ce domaine, les conditions d'une administration correcte de la justice. Nos réponses face aux crimes des personnes psychotiques resteront forcément insatisfaisantes, comme le sera peut-être notre débat d'aujourd'hui. Il est pourtant de notre responsabilité de les traduire dans des politiques publiques plus efficaces.

le jeu, permettre aux victimes de faire leur deuil et faire en sorte qu'il puisse y avoir un vrai procès, après bien des erreurs dans la conduite de cette affaire. Malheureusement, la Cour de cassation n'en a pas décidé ainsi, avec tout le respect que j'ai pour les magistrats. Ceux-ci se sont eux-mêmes légitimement

ce texte mal ficelé. J'entends bien que l'on ne légifère pas dans l'émotion, mais légiférer sur la demande des magistrats de la Cour de cassation, ce n'est pas légiférer dans l'émotion à une demande de la magistrature pour lui permettre de mieux juger. Dans ces conditions, il me paraît tout à fait normal que le législateur fasse son travail.

Il y a des familles, servez-les

tout simplement. Par conséquent, on modifie l'équilibre de notre processus judiciaire. Il faut que la chambre de l'instruction fasse son travail, ce qui n'est pas du tout exclusif

; il est seulement prévu un renvoi devant les juridictions du fond en cas de fait fautif ayant causé l'abolition temporaire du discernement. Nous n'avons donc aucune volonté de contourner les dispositions de l'article 122-1,

elle peut parfaitement se réunir en l'absence de la personne responsable de la mise en examen. En tous les cas, elle ne propose un sursis à statuer que lorsque les personnes ne sont pas en état d'être jugées.

nous souhaitons permettre au juge du fond de décider, lorsque l'origine de l'absence de discernement résulte du comportement du mis en cause, qu'un procès ait lieu, que cette absence de de discernement soit définitive ou temporaire. L'objet du présent amendement est donc de renvoyer au juge du fond le soin de statuer sur le caractère temporaire ou non de l'abolition de discernement. Quel est l'avis de la

pas plus que la non-prise d'un traitement médicamenteux consécutif à une pathologie psychiatrique qui ne serait pas imposé par une autorité judiciaire au titre d'une obligation de soins. Pour l'ensemble de ces raisons, il nous paraît indispensable de supprimer l'adjectif « fautif » de l'article 1, afin de ne pas limiter la caractérisation des cas dans lequel le comportement du mis en cause a contribué à l'abolition de son discernement, quand bien même ce comportement n'est pas constitutif, en soi, d'une infraction pénale. Tel est l'objet de cet amendement, qui nous semble essentiel pour conforter cet article. Quel

Nous avons d'ailleurs rejoint l'analyse de la commission des lois et du rapporteur afin que les familles des victimes, voire les victimes, si elles sont encore en vie, puissent bénéficier d'un procès, qui est

de La Gontrie. Nous l'avons dit, nous sommes défavorables à l'article 1 pour autant, nous proposons ici une précision procédurale procédé à l'examen de l'irresponsabilité éventuelle par la juridiction de jugement avant l'examen de l'affaire au fond.

: La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. Le discernement est nécessaire à l'établissement de l'imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l'aptitude à la sanction supposant d'en comprendre le sens. C'est pourquoi il nous est apparu utile et opportun d'inscrire dans le code pénal une définition du discernement.

C'est une piste sur laquelle je travaille et qui a nourri ma réflexion. J'ai préparé un texte qui vient d'être soumis au Conseil d'État. Pour l'instant, je vous demande donc de retirer cet amendement,

par décision motivée, être admises en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur le modèle des soins sans consentement. Le présent amendement prévoit la possibilité nouvelle pour le juge du fond, conformément à la recommandation n° 10 du rapport de la mission sur l'irresponsabilité pénale rendu en février 2021, de prononcer, en complément de cette hospitalisation, une mesure de sûreté d'obligation de soins dont la durée pourra aller jusqu'à vingt ans. De nombreuses mesures essentielles au bon fonctionnement du système judiciaire, notamment celle sur la revalorisation du travail des experts, sont d'ordre réglementaire,

Il est logique de vouloir éviter ce qui pourrait être assimilé à des sorties sèches, et de soumettre les personnes dont le discernement a été aboli, de manière temporaire ou non, à un suivi post-hospitalisation. Quel est l'avis de la commission ? La commission a donné un avis favorable à cet amendement. monsieur le ministre,

un arrêt du traitement, une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants peuvent faire partie de la maladie plutôt qu'en être la cause. Ces situations sont d'ailleurs très fréquentes dans le cas des psychoses les traitements administrés peuvent avoir des effets inhibiteurs qui minent toute activité quotidienne, de sorte qu'on peut leur substituer, à tort pour nous, mais à raison pour les patients, des toxiques qui soulagent sur le moment. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas concevable de revoir l'échelle des peines au détour d'une proposition de loi que je qualifie encore « de circonstance

les coups et blessures ayant entraîné la mort, les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'homicide involontaire et les blessures involontaires. Les dispositions prévues à cet

J'ajoute que quarante-trois femmes ont déjà été assassinées par leur conjoint depuis le début de l'année. La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société. C'est un combat universel. Un certain nombre d'associations, de parlementaires et de juristes mènent ce combat depuis plusieurs années, mais celui-ci ne progresse jamais assez vite.

Sur ce point, l'expert psychiatre a reconnu, pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France, que l'accusée était atteinte, au moment des faits, du syndrome de la femme battue. Je rappelle que le Canada reconnaît ce syndrome depuis 1990. Concrètement, la personne qui en est atteinte ne peut plus prendre de décision raisonnable et raisonnée. Toutes les attaques du conjoint violent touchent à l'intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu'elle subit. Cet état de soumission et de danger de mort permanent, vécu pendant des années, peut entraîner un comportement extrême. Cela aboutit, malheureusement, dans la plupart des cas au suicide de la victime de violences. Dans certains cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint, car il n'y a pas d'autre issue que de le tuer pour ne pas mourir : « C'est lui ou moi

impunément ces actes de barbarie. Cet amendement, déposé par notre collègue Valérie Boyer, permet d'apporter enfin une réponse à cette situation en prenant en compte la réalité des victimes qui ont traversé, en silence souvent,

L'une des raisons des divergences entre les experts ou les collèges d'experts, dans les situations où le passage à l'acte pénalement incriminé a eu dans les situations où le passage à l'acte pénalement incriminé a eu lieu sous toxiques, tient au fait que certains d'entre eux prennent en compte la position psychique du sujet au moment de la prise de la substance psychoactive pour rejeter l'atteinte au discernement, tandis que d'autres

Les experts pourraient poser la question suivante - laquelle s'inscrirait dans une nomenclature - : décrire les conditions, les motivations et les conséquences, dans l'hypothèse où des circonstances telles que la prise de toxiques ou un arrêt d'un traitement médical peuvent avoir provoqué ou accentué un état pathologique altérant ou abolissant le discernement, entravant ou abolissant le contrôle des actes. Tel est l'objet de cet amendement.

de garde à vue à la seule compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure, en excluant expressément les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire.

de vote. Je suis, comme tous les membres de mon groupe, bien conscient du trouble, de l'émoi, de la colère exprimés par les personnes qui ont trop souvent l'impression que l'irresponsabilité pénale signifie que le mis en cause échappe à la justice. Aussi violent que cela puisse paraître, tel n'est pas le cas : la justice s'intéresse aux faits et, lors d'une audience contradictoire qui peut durer des heures, où la parole est donnée aux victimes et aux parties civiles, elle se prononce sur la responsabilité du mis en cause. Il convient également de rappeler que l'irresponsabilité pénale ne signifie pas que l'individu déclaré irresponsable sera remis en liberté : il est placé en hospitalisation sous contrainte et des mesures de sûreté, pouvant aller jusqu'à 20 ans, peuvent être prononcées à son égard. Ces mesures, en plus de soigner l'individu, ont pour objet d'évaluer sa dangerosité et d'empêcher la récidive. Je crains qu'en l'état cette proposition de loi ne puisse améliorer la situation, et l'amendement retenu à l'article 1

Aujourd'hui, notre système judiciaire fonctionne. Certains juges, s'appuyant sur des expertises, ont déjà retenu la responsabilité de personnes, qui, du fait de l'ingestion d'alcool ou de stupéfiants, plaidaient l'irresponsabilité. C'est pourquoi, soucieux de préserver l'équilibre de l'article 122-1 du code pénal, de renouveler notre confiance dans la capacité des juges à évaluer l'abolition du discernement des mis en cause en s'appuyant sur les expertises psychiatriques, et prudent quant à la possibilité pratique de se prononcer sur un fait

une bipartition entre, premièrement, l'examen de l'irresponsabilité éventuelle, et, deuxièmement, l'examen au fond par la juridiction du fond,